pour 2023 dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 15 ah. Je mets d'ailleurs tout de suite aux voix, l'article 15 ah. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté. Amendement après l'article 15 le 1000 Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, les établissements publics territoriaux de bassin, ce sont des outils essentiels pour la gestion équilibrée et durable de l'eau, tout en développant les solidarités à l'échelle des bassins versants opérationnel l'analyse financière de ces établissements montre une fragilité pour assurer leur mission dont notamment celles relatives à l'expertise à la planification à la programmation territorial avec l'ensemble des des acteurs, ce qui est particulièrement essentielle dans le contexte d'adaptation au dérèglement climatique, les décisions territoriales doivent s'appuyer sur une connaissance fine des fonctionnement des écosystèmes des fonctionnement hydraulique et sur une animation territoriale pour associer l'ensemble des parties prenantes et construire co-construire les plans d'action, vous le savez, toutes les collectivités locales, quelle que soit leur localisation, leur richesse doivent aussi pouvoir être accompagné sur ces questions de gestion intégrée de l'eau par bassins et notamment pour l'exercice de la compétence Gemapi d'une part mais aussi pour les missions relatives à la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, les financements pour l'ingénierie sont aujourd'hui de plus en plus complexes à mobiliser ni car il n'existe pas de compétences et de recettes fléchés, il est indispensable que les EPTB bénéficie d'un auto-financement pérenne pour assurer leur mission socle qui sont inscrites dans l'article Haddock les concernant et donc d'une recette fléchés, la majoration de la redevance prélevée levée par les agences de l'eau prévu de par l'article L 213 tiré 10 tiré 9 du code de l'environnement pour la mise en oeuvre des sages pour les EPTB, n'a jamais pu être mobilisés malgré plusieurs dossiers qui ont été déposés en ce sens, plusieurs freins ont été identifiés, dont la mise en place du plafond, mordant des recettes des agences de l'eau et le manque de précision du texte, entraînant des interprétations différentes, il est proposé, donc de mettre en place une disposition plus simple visant à mettre en oeuvre une recette fléchés pour les projets portés par les EPTB, constitué d'une majoration de 3 à 10 % des redevances levée par les agences de l'eau cette recette n'est pas affectée aux agences de l'eau et non pas intégré dans le plafond, mordant. Merci, cher collègue, avis de la commission sur le rapporteur. C'est une demande de retrait en fait par votre amendement, vous attirez légitimement. Notre attention sur le sujet du financement effectivement de programme j'ai Mappy de programmes de protection des territoires. Pour des les inondations mais pas seulement, et vous l'avez dit, et le financement par les agences de l'eau avec ce fameux plafond mordant, il y a plusieurs éléments de réponse en tous les cas pour cette année deux notamment le l'annonce de la première ministre qui propose de libérer 100 millions d'euros sur finalement une forme de déplafonnement à hauteur de 100 millions d'euros en relâchant la trésorerie des agences de l'eau et puis ce que nous avons également obtenu par ailleurs dans le PLFR mais je pense qu'il faut être attentif à cette question du financement qui n'a jamais finalement été bien prévus par le transfert des compétences dans les territoires et pour les EPTB, ça met d'ailleurs en tension, les financements des collectivités territoriales, parce que quand on est sur un EPTB, on est bien souvent sur un périmètre plus large que une, 2 ou 3 intercommunalité, donc je pense que c'est un peu le périmètre concerné, si l'on veut mener les les projets et les programmes imaginez est nécessaire pour mettre les populations et les acteurs économiques également dans des situations de sécurité, on a un vrai problème de ressources, une demande de retrait mais je devine que le ministre, il va nous donner en plus peut-être de bonnes nouvelles sur des moyens supplémentaires. De très bonne nouvelle, monsieur le rapporteur général, moi je veux insister sur plusieurs éléments dès cet été, la première ministre a annoncé un 1er relèvement du plafond de dépenses des agences de l'eau de 100 millions d'euros. Il y a quelques semaines, elle a annoncé un place un relèvement supplémentaire du plafond des agences de l'eau de 100 millions d'euros, je vous rappelle qu'elle bénéficie d'une taxe affectée, elles ont un plafond de dépenses et dans le cadre du PLFR du projet de loi de finances rectificative, vous avez adopté ici un amendement qui a été conservé dans le cadre de la commission mixte paritaire, le texte ayant été adopté hier à l'Assemblée nationale de la CNP, il sera adopté, j'espère, demain, ici au Sénat, qui prévoit, et c'était une initiative du rapporteur général Husson 50 millions d'euros de crédits supplémentaires pour les agences de l'eau, vous voyez, donc il y a un investissement massif supplémentaire en cette année 2022, c'est un enjeu essentiel évidemment pour l'entretien du réseau pour l'investissement et pour la prévention, notamment vis-à-vis des sécheresses, et donc on est au rendez-vous, collectivement, pour répondre aux besoins de financement des agences de l'eau. Bien Monsieur Gillet, l'amendement est maintenu Monsieur le rapporteur, l'amendement est maintenu, parce que si ces bonnes nouvelles en direction des agences de l'eau effectivement sont confirmées, il y a donc aucune difficulté pour répondre à à demande puisque la demande c'est de flécher des crédits en direction des EPTB donc on a les moyens de pouvoir le faire, donc en l'occurrence je maintiens cet amendement. Bien donc maintien de de l'amendement, donc avec un double avis défavorable, je le mets aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous passons à l'article 15 mai et j'ai une demande de prise de parole de Madame avait. Merci monsieur le président, l'idée de cet article et de mettre en place un Loto de la biodiversité et ainsi créer un jeu de grattage mission biodiversité à l'instar du Loto mission Patrimoine cet article s'inscrit dans une volonté de valoriser la protection de la biodiversité, ce nouveau jeu de grattage, permettrait de dégager une source supplémentaire de financement de l'ordre de 10 millions d'euros la première année d'exploitation de jeu en faveur de la biodiversité, le montant collecté permettrait de soutenir des projets en faveur de la préservation et la restauration de la biodiversité dans les territoires, en sensibilisant et associant les Français à cette cause à laquelle ils sont très attachés, c'est la 2ème cause de préoccupations des Français après le pouvoir d'achat alors lors du séminaire du lancement de l'en février 2020, le président de la République avait réaffirmé son ambition d'accélérer notre politique de protection de la biodiversité, cet article est un des moyens d'y parvenir en considérant, il n'y a pas de raison de ne pas mettre sur un même pied d'égalité, la valorisation de notre Patrimoine et le soutien de notre Patrimoine culturel, pardon et la préservation de notre environnement, je soutiens pleinement le maintien de cet article et je voterai contre sa suppression, je vous remercie. Merci madame avait donc maintenant nous avons 3 amendements identiques de suppression, le 1er présentée par Madame Lavarde. Oui, merci Monsieur le Président, alors c'est parfait, je vais pouvoir répondre à notre collègue qui vient en renfort mais attendez, vous nous dites ce Loto de la biodiversité va venir financer des actions est-ce que vous connaissez le rendement attendu de la mesure 10 millions d'euros, 10 millions d'euros, donc c'est pas avec ça qu'on va financer la biodiversité, l'idée derrière c'est soit à devenir créer un nouveau jeu pour la Française des Jeux, soit devenir financer des actions de communication pour parler de la biodiversité, alors je trouve que c'est à ce moment-là, tout ce qui est fait par le ministère par l'OSB par les collectivités par tout un tas de personnes qui prône, matin, midi et soir, qu'effectivement l'enjeu climatique est un vrai sujet et je pense que le faire par un Loto c'est dangereux, c'est même un enjeu de santé publique, il vous a pas tout s'est échappé que le gouvernement, par un autre ministère, celui des Affaires sociales,

un amendement qui vient créer un nouveau jeu et enfin juste peut être je j'avoue que j'étais assez choqué de recevoir une invitation du directeur général de l'Office national de la biodiversité qui m'invitent à un déjeuner débat sur l'engagement des entreprises pour la préservation de la biodiversité avec un témoignage Stéphane Pallez, présidente-directrice générale de la Française des Jeux. mes propos vont s'inscrire complètement dans les propos qui viennent d'être tenus par Christine Lavarde j'ai envie de dire un moment puisque j'ai compris que c'était d'abord une initiative d'un député Renaissance, le débat n'ayant pas eu lieu à l'Assemblée nationale, on nous le met dans le texte, à un moment donné, je voudrais qu'il y a un moment de vérité. 10 millions d'euros pour faire de la com. Alors qu'il y a un loto. Spécifiques. Qui est sur le Patrimoine. Il est finalement assez bien identifiés, il a, me semble-t-il, celui-ci a un Avantage, c'est qu'il permet de donner un coup de projecteur sur un certain nombre de biens patrimoniaux et qui reflètent l'identité de la France. Mais là on touche à des missions régaliennes de l'État, on est sur le sujet de l'écologie au sens large et de la biodiversité qui mérite bien d'autres moyens, alors c'est beau d'avoir un budget vers c'est beau d'expliquer à longueur de temps et de conférences, d'aller à la COP27 pour aussi peu de résultats et aller chercher l'addiction possible au jeu comme ça vient d'être dit, alors que le ministère des Affaires sociales, que tout le monde se met comment dirais-je, au diapason pour essayer de mettre en place, dispositif pour lutter contre les jeux de hasard, mettons une politique des politiques communes et articulé, sous l'autorité de l'État avec les territoires également avec les acteurs privés parce que cette affaire-là, c'est une affaire commune partagée qui concerne aussi bien les entreprises l'État que nos concitoyens, mais de grâce, tournons le dos à ce que j'appelle un vent de populisme Vert qui ne me paraît pas acceptable en tous les cas, que ce soit soutenu par l'État, dans ces conditions, notre démocratie est le sujet sont trop importantes pour laisser aux mains de jeux de hasard, vraiment, de mon point de vue cet irresponsable. madame Préville. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc je suis dans la lignée de ce qui vient d'être dit et je reprendrais ce que les auteurs de cette proposition ont exprimé à l'Assemblée nationale pour faire passer par amendement, ce jeu de grattage, consacré à la biodiversité, comme vous l'avez compris, il s'agirait d'une manière innovante et engageante d'impliquer les citoyens alors innovation bien sûr, le mot est lâché ce mot qui a dynamité l'idée même de progrès le l'habiller également 2 engageant d'impliquer les citoyens, voilà une proposition mauvaise proposition provision pernicieuse, très bien habillé, je, je dirais, en en gros les mêmes choses à une autre, une partie du financement de la diversité ne peut pas reposer sur un jeu de hasard la biodiversité me mérite des ressources pérennes à la hauteur de l'enjeu que représente sa protection, cela ne peut s'appuyer sur une incitation aux jeux d'argent, j'ai moi-même déposé au PLFSS des mesures de taxation sur les jeux d'argent en ligne, les jeux d'argent sont source de comportements addictifs, ils exposent les personnes non seulement à des difficultés sociales et financières, ce qui est, de fait, mais aussi à des problèmes psychologiques, on parle d'addiction dans l'acceptation totale du terme, c'est-à-dire une spirale infernale et l'enfer pour les familles qui le subissent, c'est également bon à donner un bon prétexte pour jouer, il s'agit de Green washing du jeu, je ne peux pas m'inscrire là-dedans, le mélange des genres, jeux d'argent biodiversité est très discutable, je le dis, que je me comme je le pense et éthiquement c'est rédhibitoire, c'est le télescopage d'idées qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, l'habit de biodiversité et l'enjeu de notre survie et ce n'est pas un petit sujet à de notre survie et d'ailleurs à pas si long terme que cela enrayer la baisse de biodiversité relève d'une politique de long terme et sûrement pas de cette façon-là, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre.

est une des conséquences de l'effondrement des écosystèmes et de la façon dont on les malmène donc proposer face à cet enjeu immense qu'est la préservation du vivant, le rétablissement d'écosystème de faire un loto de la biodiversité, je n'insiste pas sur le caractère dramatique de l'addiction au jeu, mon collègue de Sud ailleurs il reviendra, je veux juste dire que le vivant mérite beaucoup plus que les 10 millions que ce Loto pourrait rapporter et même que les 30 les 30 millions du fonds pour la biodiversité, il mériterait une inflexion de la plupart de nos politiques publiques et à l'évidence, nous ne voterons pas cette proposition. Allez-y, chers collègues. du réchauffement climatique sous l'angle de l'auto, ça quand même paraître dérisoires et je pense que le mutisme du de Monsieur le Ministre, par rapport à cette situation, dénote bien qu'aime l'embarras de trouver des moyens sous couvert de de bricolage et et dans une certaine mesure, un dispositif baroque pour traiter les questions de biodiversité, alors que l'ESB soit favorable en dépit du rendement ridicule que que cela comporte, je peux le comprendre, mais moi j'aurais voulu que le ministre-clarifie sa position. Merci donc nous avons un avis défavorable du ministre, il l'a donné, nous allons nous allons voter donc sur ces trois amendements identiques de suppression qui est pour.

Merci Monsieur le Président, donc c'est c'est un amendement qui vise à instaurer un prélèvement sur les jeux de casino en ligne, bien que la France soit le dernier pays d'Europe continentale à à en interdire la pratique l'offre illégale de casino en ligne et hélas plus plus plus pléthorique que jamais, or le maintien de la non-régulation des casinos en ligne constitue en fait un facteur majeur de risque pour les particuliers, mais aussi à un manque à gagner colossal pour le Trésor public, selon les dernières projections le marché illégal représenterait 1,1 milliard d'euros de produit brut des jeux, soit plus de 600 millions d'euros de recettes fiscales annuellement perdu pour l'État pour remédier à cette situation et et protéger les les 2 millions de Français fréquentant cette offre illégale, cet amendement propose donc d'encadrer la pratique des de casino en ligne tout en là, pardon assujettissement à un double prélèvement sur le chiffre d'affaires ou pour du brut des jeux merci. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur. J'attire l'attention de notre collègue sur le fait que cet amendement comporte des effets de beurre et notamment celui d'autoriser finalement indirectement les casinos en ligne, je rappelle qu'aujourd'hui seuls les jeux de cercle en ligne sont autorisés, ce qui n'est pas le cas des machines à sous et des jeux de table, la loi de finances ne me paraît pas être le moment le plus approprié pour ouvrir ce débat c'est une un avis défavorable. Monsieur le Ministre. monsieur le Président, oui, je veux dire, Monsieur le Sénateur, Rambo, que c'est une vraie préoccupation que vous soulevez, qui est celle du développement des jeux de casino en ligne et d'une offre illégale, c'est évidemment un risque pour l'addiction au jeux, notamment des plus jeunes, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux et d'ailleurs, j'ai rencontré récemment la présidente de la, de l'Autorité nationale des jeux qui va lancer une étude sur l'offre illégale et une fois cette évaluation terminée, nous envisagerons des solutions supplémentaires pour assécher cette offre illégale, donc c'est une demande de retrait dans l'attente pour cet amendement mais vous voyez bien qu'on prend le sujet très au sérieux et que nous avons l'intention d'agir sur le sujet.

Merci monsieur le président, on va parler de paris sportifs, ça a été dit par ma collègue, c'est aussi un problème de santé publique, face à un modèle très cynique, c'est un un problème de santé publique sur la loterie, on a parlé des addictions, mais sur les paris sportifs, c'est 5 à 6 fois plus addictifs que ça ça que et on a, sur un modèle économique extrêmement cynique parce qu'autant la loterie, on peut dire que c'est une forme d'impôt sur les mauvais en maths, autant là, on est sur un modèle qui va cibler les plus jeunes qui va cibler les quartiers populaires, un jeune sur 3 et je parle de jeunes de 15 à 17 ans, a déjà joué à déjà parié ça touche un tiers des jeunes de 18 à 24 ans. Aussi et donc, cet amendement vise à augmenter la taxe sur les paris sportifs en ligne cette taxe avec viendrait abonder le budget de l'Agence nationale du sport, il s'agit d'envoyer un signal, comme le dit souvent, le ministre-au monde économique pour faire le tri entre les modèles économiques toxiques et les autres, donc on propose de de passer le taux de 10,6 % à un taux de 15,9 % je vous remercie. des opérateurs de paris enregistrent des chiffres d'affaires absolument historique d'ailleurs, ça c'est constaté en en 2021 au moment des de la pandémie les médecin addictologue constate un mouvement parallèle dans leur consultation, un psychiatre qui est président de la Fédération addiction commande dans ces termes ceux qui sont visés sont les jeunes précaires des quartiers effectivement notre collègue là dit qui cherche à un avenir heureux car ceux qui sont visés sont ceux pour qui le coût de la vie par contre ceux ceux pour qui le coup sur selon Santé publique France 60 % du chiffre d'affaire des paris sportifs vient de joueurs problématiques entre guillemets dont 24,8 pour 100 de jeu excessif, donc même destination pour ces fonds augmentation donc du taux de prélèvements de d'ici ça très 6 et qui serait affectés à l'Agence nationale du sport pour développer les pratiques sportives. Merci, monsieur le rapporteur sur ces deux amendements. les les paris sportifs avec donc une question sur l'impact que ça peut avoir su cette activité, d'où la demande de David du gouvernement. Merci monsieur le président, l'objet de cet amendement si je lis l'exposé sommaire, c'est de relever cette fiscalité sur les paris sportifs pour abonder le budget de l'Agence nationale du sport, sauf que l'amendement que vous proposez est inopérant, de ce point de vue-là il ne permettra pas d'abonder les Budgets de l'Agence nationale du sport parce que si vous relevez la fiscalité vous augmentez la le taux de fiscalité, vous ne relevait pas dans le même temps, le plafond de la taxe affectée et donc ce relèvement de la fiscalité ne bénéficierait pas à l'Agence nationale du sport puisqu'il faut dans le même temps, relever le plafond de la taxe affectée pour que les ressources supplémentaires soient affectés à l'Agence nationale du sport, moi je veux insister sur le fait que dans ce PLF 2023, on prévoit une augmentation assez significative du budget de l'Agence nationale du sport puisqu'il y a 1 19 4 millions d'euros de crédits supplémentaires, ce qui porte le budget en 2023, de l'Agence nationale du sport à 265 millions d'euros, donc avis défavorable. Monsieur le rapporteur, après l'avis du gouvernement, votre avis. Défavorable, donc il y a un double avis défavorable sur ces deux amendements pas d'explication de vote Monsieur Breuiller. j'entends la la remarque de Monsieur le Ministre, qui est soucieux du des fonds à l'Agence nationale du sport les les amendements visait surtout à dire que, au fond, ces paris sportifs sont quand même quelque chose qui mérite d'être taxé plus fortement, et surtout d'être découragé mais Monsieur le Ministre, si ça ne va pas à l'Agence nationale du sport, ça ira dans les caisses de l'État et j'ai cru comprendre que ses caisses étaient singulièrement dégarni, donc vous pouvez donner un avis favorable, c'est une recette je je ne comprends pas que vous refusiez une recette pour les caisses de l'État. Bien, nous allons passer donc on voit sur ces deux amendements qui est favorable. Enfin au premier puisqu'ils ne sont pas exactement identique, donc il est favorable au premier. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, donc le 2ème tombe, nous passons à l'Arctique

Donc Monsieur dessus pour le premier amendement 904. Merci monsieur le président, c'est évidemment vu le le le montant un amendement d'appel j'ai bien entendu la défense de chacun, de la biodiversité et à quel point il fallait avoir de l'ambition sur la protection de la biodiversité, on a fait cet amendement pour appeler à remettre à plat toute notre modèle de vision de l'aménagement du territoire, notamment ceux qui concerne les transports, puisqu'il s'agit de de d'interpeller sur le développement de projets routiers actuellement, on a recensé 55 projets routiers dans les dans les cartons de l'État pour 18 milliards d'euros, ces projets ne sont plus à la hauteur de l'enjeu à la fois climatique mais aussi de protection de la biodiversité, puisqu'il bétonne un certain nombre d'espaces naturels ou agricoles et donc nous souhaitons interpeller un peu l'état à ce sujet, pour remettre à plat et proposer d'autres développements. Du des, des modes de déplacement, on l'a bien vu que des des modes de déplacement, otages de la voiture individuelle, c'est-à-dire en développement du routier et que du routier, hé bien, nous arrivons à parfois quand il y a des coups sur la le le sur l'énergie à une hausse des coûts sur l'énergie à devoir renflouer à devoir soutenir un modèle de développement qui ne nous convient pas, donc nous proposons un amendement d'appel évidemment. Je le rapporteur. Demande de retrait Monsieur le Ministre, même avis double demande de retrait. Il est retiré ensuite trois trois amendements qui font l'objet d'une discussion commune le premier

qui, en 1999 a institué le fait de faire des ponctions des des recettes des agences de l'eau pour alimenter le budget de l'État, c'est toujours intéressant de de se rappeler un petit peu de ce qui s'est passé, voilà quelques années, c'était en 99 à l'époque, on voulait faire de de l'écologie, mais en même temps, c'était déjà lui en même temps, vous voyez, ça a commencé déjà là et aujourd'hui on a institué le ce qu'on appelle le plafond mordant, alors c'est peut-être un peu mieux mais c'est pas du tout satisfaisant puisque ça plafonne les les financements pour les agences de l'eau et ça limite les capacités d'action des agences, alors même qu'on leur demande de plus en plus de d'actions à mener en leur demande de faire en sorte que les adductions d'eau soit moins fuyantes, on leur a mis le l'OSB à financer ces 400 millions d'euros, si on veut faire des travaux pour améliorer la performance des adductions d'eau, c'est 200 millions d'euros par an qu'il faudrait remettre et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, hé bien il y a pas suffisamment de financements dans les agences de l'eau, donc on va chercher des financements à la DETR pour les collectivités pour qu'il puisse financer leurs opérations alors c'est complètement ridicule, alors que c'est à l'agence de l'eau, de financer, donc moi je vous propose de rehausser ce plafond mordant parce que l'eau doit payer l'eau c'est la la règle donc moi je suis d'accord pour alors on m'a dit qu'il était favorable cet amendement mais qu'il fallait que je le rectifie moi je veux bien mettre le plafond mordant à la hauteur de ce qui est prévu pour qu'on puisse avoir une satisfaction sur cet amendement. Merci, cher collègue, ensuite, 2 amendements identiques Monsieur Bonhomme, le premier. monsieur le président, oui, mais dans le même esprit, effectivement, que que celui de mon collègue Pointereau trop, il s'agit de de déplafonner le fameux plafond mordant qui vient grever les capacités d'intervention des agences de l'eau et depuis de nombreuses années, donc là vous savez c'est un truc que je de raisonnable le plafonne à à 2 milliards 300 je voudrais dire que nous sommes le onzième programme et que, d'ores et déjà au niveau de l'espèce, l'Agence Adour-Garonne pour ce qui nous concerne, nous voyons les effets défavorables, puisque à la fois on a développé l'émission et le Champ d'intervention des agences ah émeutes, hein, on a depuis de nombreuses années, institué le plafond mordant et je rappelle même que pour les années à partir de 2013, 2014, de mémoire, au motif qu'il y avait de la trésorerie importante des agences, on a déjà ponctionné, donc ça fait plusieurs milliards d'euros qui ont été détournées en quelque sorte de la mission première fixé par les redevances que touchent les agences et aujourd'hui, avec un effet retard on on voit les effets l'assainissement collectif l'assainissement non collectif, l'émission qui soit élargi, on voit que le onzième programme a été revu à la baisse à peu près partout et le 2ème programme qui est en cours de discussion va dans les mêmes dans le même sens, donc je voudrais dire que comme notre collègue Pointereau là, l'a déjà dit dans d'autres débats, la loi de 2005, elle a notablement été piétinés, voilà l'eau paye l'eau, ça fait bien longtemps que l'eau ne paye plus l'eau, c'est l'eau paye là les déficits de l'État et la difficulté et la l'incapacité de l'État a qui Bresson, budget. merci Monsieur Gillet amendements identiques. Merci monsieur le président, pas tout à fait puisque lui, il vise à la suppression du plafond mordant, même si vous propose de le rehausser à 2 8 milliards d'euros la suppression et en même temps, il faut mettre en perspective le fait que il est nécessaire, il serait nécessaire de mettre en place au niveau national, Monsieur le Ministre, une forme de caisse de solidarité interbassins qui permettrait de solidarité entre les agences de l'eau en fonction de projets à caractère particulièrement structurants, je voudrais insister sur un des sujets sur le financement de la Gemapi, et plus particulièrement de la prévention et la protection contre les inondations, il y a une énorme différence entre des petits cours d'eau et des cours d'eau majeur et sur les cours d'eau majeur, il y a une grande difficulté pour financer la prévention sur les inondations, même si l'intervention de l'État, aujourd'hui elle est de l'Ordre de 30 % au maximum et les collectivités de peuvent pas suivre par rapport à ça, or les agences de l'eau, les programmes des agences de l'eau sont très modeste, puisqu'ils n'interviennent que sur les études et on n'accompagne pas les collectivités à ce niveau-là, le fait de déplafonner aujourd'hui permettraient une solidarité aussi interbassins et d'intervenir aussi plus directement sur des ouvrages particulièrement coûteux, donc voilà je souhaite maintenir bien sûr cet amendement, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Un avis favorable pour relever le plafond à hauteur de 2 milliards trois je crois que les moyens, ça a été dit à la fois par les auteurs des amendements mais j'ai eu l'occasion de je pense surtout que, avec le relèvement du plafond, c'est aussi finalement une incitation à l'endroit du gouvernement pour augmenter les ressources des agences de l'eau. J'ai entendu et compris dans cette enceinte, parfois, des critiques assez virulentes à l'endroit des agences de l'eau, parce que les élus ont le sentiment que pour une part le, comment dirais-je, leur faculté d'intervention n'est pas en lien Direct, je veux juste te dire que cette les agences de l'eau, c'est plutôt une une des enceintes dans lesquelles sont mêlés, tous les acteurs, les acteurs de l'État, le monde agricole, les industriels et les élus, c'est donc quelque part à un parlement de l'eau ou à la fois il y a des débats importants sur les orientations et dans les 6 agences de bassin ces débats donne lieu à des orientations. Adapté au territoire, c'est vrai, on l'a vu tout à l'heure pour par exemple les EPTB, les démarches également autour des actions de biodiversité, puisque, comme ça a été rappelé cette aujourd'hui aussi l'eau qui finance des actions de biodiversité, il a finalement une logique donc avis favorable et effectivement je j'ai entendu le sénateur Pointereau dans son propos liminaire, dire qu'il était prêt à rejoindre, me semble-t-il, et ce serait la condition, effectivement, d'être également favorables à son amendement. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, la gestion et la protection de la ressource en eau est une priorité du gouvernement et nous avons pris un certain nombre de mesures pour soutenir les investissements des agences se sont par ailleurs des sujets qui sont intégrés au secrétariat général à la planification écologique rattaché à la première ministre avec un chantier spécifique dédié à l'eau et à l'optimisation de la ressource en eau et à son financement je suis défavorable à l'amendement qui est proposé à cette disposition, pour plusieurs raisons. D'abord parce que rehausser surtout dans ces niveaux-là, le plafond des taxes affectées aux agences de l'eau se traduirait in fine et par une augmentation de la fiscalité sur l'eau qui toucherait le contribuable les agriculteurs et les entreprises puisque l'écrêtement de la taxe affectée l'an dernier, reverser à l'État, c'est au tour de 20 millions d'euros si vous rehausser le plafond à hauteur de 400 millions d'euros, soit vous relever la fiscalité pour pouvoir financer ce relèvement et donc ça peut toucher les consommateurs, les agriculteurs, soit vous ne le relever pas et à ce moment-là, ça veut dire que vous allez prendre des fractions de taxe affectée qui vont à d'autres organismes, il y a l'Office français de la biodiversité, je crois, et d'autres donc pour ce 1er sujet défavorable, l'autre raison, c'est que ce mécanisme de plafonnement permet aux agences de l'eau, de disposer de ressources importantes, ça a été dit leur trésorerie a augmenté de 370 millions d'euros en 2018 à environ 700 millions d'euros aujourd'hui et je veux redire que pour leur permettre d'investir pour leur permettre de dépenser cette trésorerie, la première ministre a annoncé de relèvement du plafond de dépenses cet été un en 1er relèvement de 100 millions d'euros il y a une semaine ou 10 jours, un second relèvement de 100 millions d'euros et qu'à l'initiative du rapporteur général dans le PLFR vous avez adopté, il est dans le texte de la CMP, un amendement qui prévoit 50 millions d'euros de crédits supplémentaires, j'ajoute enfin que le fond Vert permettra également de soutenir les actions des agences de l'eau, notamment outre-mer et en faveur de la biodiversité. Merci, monsieur le Ministre, donc un amendement favorable de la commission sur les deux amendements qui porte le plafond à 2 milliards 300 millions d'un amendement défavorable du gouvernement Monsieur Pointereau est ce que vous voulez rectifier votre amendement. oui, merci Monsieur le Président, moi j'ai l'impression que le Fonds Vert il va depuis hier, c'est plus, c'est plus de milliards qu'il faut, c'est 10 milliards, hein, parce que vous l'avez mis à toutes les sauces non mais moi je comprends pas Monsieur le Ministre vous annoncer que de madame la première ministre a débloqué 100 millions d'euros, plus 100 millions d'euros, plus 50 millions d'euros, ça fait 250 millions d'euros, et moi je et vous voulez pas qu'on a qu'on augmente le plafond mordant mais c'est c'est pas logique, c'est pas cohérent ce que vous nous dites, moi je veux bien, si vous voulez 2 milliards 300 millions d'euros pour qu'on soit en cohérence et que ça soit un 1er pas pour pour l'année prochaine parce que il y a un vrai besoin dans nos agences de l'eau, de faire du du financement, le l'OSB qu'on a mis une compétence supplémentaire aux agences de l'eau, c'est 400 millions d'euros par an 400 millions d'euros on veut diminuer les les fuites sur nos réseaux, un milliard de mètres cubes d'eau perdue en France c'est 1000 bassine, messieurs, mesdames, messieurs les mes collègues écologistes, donc il faut il faut qu'on ne on arrive aujourd'hui à mettre des moyens supplémentaires, sans pour autant augmenter la la fiscalité parce qu'on est quand même pas non plus fou à ce point là d'augmenter la fiscalité de de l'eau dans nos dans nos territoires, on est quand même de trop proche des territoires pour faire des des bêtises pareilles, donc voilà, moi je souhaite le mettre 2 2 milliards 300 millions d'euros pour qu'on puisse être en cohérence avec mon collègue François Bonhomme. Bien, donc on a trois amendements identiques, j'ai plusieurs demandes de prise de parole, mais avant, monsieur le président de la commission des finances Claude Raynal. je vais essayer, mes chers collègues, de vous convaincre de pas trop faire de défense voilà de trop intervenir sur article parce que Zora Arctique et sur amendement, je vous signale que depuis jeudi, on essaye de faire rentrer 1700 amendements dans un verre qui permet pas de le faire rentrer que ce matin, on y est presque et que maintenant on y est plus, très simplement, donc je voudrais vous rappeler des souhait d'échouer le souhait ses interventions pour présenter l'amendement pas plus d'une minute le règlement vous donne deux minutes vous appréciez mais pas plus d'une minute, si possible pas trop de relance et pas trop d'avis personnel, en m'excusant parce que on a envie tous de participer à des débats comme celui-là, par exemple, mais à la sortie, je vous indique qu'à 13 heures, ça veut dire la chose suivante : ça veut dire qu'on n'aura pas fini, ça veut dire que si on n'a pas fini à quatorze heures trente on ne peut pas voter sur les recettes, ça veut dire que nos collègues et peut être même ici certains quand déjà prévu un train, un avion à quinze heures c'est même pas la peine, vous pouvez déjà tout annuler, je vous le dis, et c'est pas respectueux, voilà il faut respecter le travail qui a été fait depuis jeudi, qui nous a amenés à être à peu près dans les temps, donc soyons dans détend essayant à 13 heures sinon aussi toute l'émission, qui est comment se sont renvoyés, donc voilà, attention à ce qu'on fait, je crois qu'il faut savoir tout simplement, tranquillement, écoutez la position du ministre ou pas trop le relancer, de toute façon, les positions de votre et d'une certaine façon, en m'excusant plus par le rapporteur général que par le ministre ici dans cette assemblée, donc, de grâce, voilà pression comme ça j'aurais prévenu mais après la responsabilité est la vôtre, merci. Donc je vais respecter les demandes de prise de parole, mais chacun agira en responsabilité, comme l'a dit le président, donc Monsieur Gremillet. Oui merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. C'est quand même un sujet, moi, je voudrais remercier de poser la position de notre rapporteur général je soutiens ces amendements pour 3 raisons. La première, n'oublions pas qu'aujourd'hui on aurait on a quand même du mal de regarder tous les Français dans les yeux pour celles et ceux qui ne sont pas à l'assainissement collectif à individuel, on les a bien abandonner complètement au en plein milieu du gué, c'est qu'à le dire, deuxièmement. Monsieur le Ministre. Effectivement, on a un sujet sur l'eau, aujourd'hui il y a des investissements énormes pour permettre effectivement que le cycle de l'eau sortie de la station d'épuration puisse à nouveau réalimenté réalimenté ce sont des investissements qui concerne à la fois les collectivités à la fois les entreprises énorme et puis dernière remarque, Monsieur le Ministre le Front Vert. ce sont quand même des moyens qui proviennent du contribuable, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel donc aujourd'hui ne m'mentons pas français permettant effectivement que l'argent qui provient de l'ensemble des ménages, des entreprises pour financer l'eau reste effectivement l'eau donc je soutiens vraiment ces amendements, ils sont essentiels pour, effectivement, été au rendez-vous. Merci monsieur le Président, rassurez-vous, je serai bref mais enfin le Parlement, il est là pour parlementer, il est pas là seulement pour voter, hein, je soutiendrai aussi évidemment les les amendements de mes collègues, parce que c'est bien beau d'avoir des discours écologique vertueux, faut avoir une stratégie vertueuse et c'est vrai, comme l'a souligné Rémy Pointereau c'est totalement incohérent d'aller rajouter un petit peu de sous pour les ARS, alors qu'on les deux pour les agences de l'eau, pardon, alors qu'on les ponctionne et comme l'a dit Daniel Gremillet, moi je suis dans un département où il y a énormément de communes qui doivent interrompre des projets ou ne pas faire aboutir des projets d'assainissement collectif, voire même. De révision d'assainissement non collectif, parce que les agences de l'eau, il y en a deux sur mon territoire Seine Normandie Artois Picardie ne peuvent plus financer, donc il faut rendre ces moyens qu'on là aux agences de l'eau et tout ira mieux. mon expression vise justement à donner le sens du vote et par rapport à l'intervention du président de la commission des finances, je pense que ça peut avoir un intérêt puisque nous voterons favorablement à l'amendement rectifier de de Monsieur Pointereau et il devrait donc faire tomber nos amendements, donc je voudrais préciser que. Par rapport aux disponibilités financières des agences de l'eau, si les agences de long des dispositifs financière, il faut à ce moment-là que les réglementations d'intervention soit modifiée pour permettre d'intervenir, notamment sur des programmes de prévention et de protection contre les inondations, à l'heure actuelle, les agences de l'eau n'interviennent pas sur les politiques d'investissement à ce niveau-là, donc, s'il dit la la l'argent disponible, allons-y, à l'heure actuelle, il y a des communautés de communes qui n'arrive pas à financer leurs ouvrages sur la prévention des inondations. Merci Monsieur bonhomme. Oui, en une minute, monsieur le président, moi, dans le même sens, d'abord je voudrais dire que on a été quand même raisonnable de 2 milliards trois c'est surtout pour rompre avec une pratique qui dure depuis des années, ce qui a été dit par mes collègues, effectivement, je confirme, il y a beaucoup de reports de projets, il y a beaucoup, même d'annulation de proches, je connais des petites communes qui, depuis des années, préparer l'assainissement de leur collectif et qui ont dû renoncer purement et simplement

donc on a vraiment les conséquences sous les yeux de de plusieurs années de de pratique et puis ensuite, Monsieur le Ministre le fond Vert, cessez de nous dire à chaque fois qu'il y a un problème ou une question de sortir la martingale le fond Vert, faudrait pas quand même que le fond Vert devienne le cache-sexe de votre nom politique a maintenu, rien à dire, en

elles, ont un plafond sur leurs dépenses parce qu'elles ont le droit de dépenser et ensuite il y a un plafond sur la taxe affectée aujourd'hui, elles ont, j'ai donné le chiffre tout à l'heure, je crois, 700 millions d'euros de trésorerie, ça a beaucoup augmenté et donc l'important pour qu'elle puisse investir et dépenser cet argent, c'est moins le plafond des taxes affectées qui de toute façon, et au maximum, il y a 20 millions qui est créé pour l'État que le plafond de dépenses pour leur permettre de dépenser la trésorerie qu'elles ont, on a annoncé de relèvements cette année de 100 millions d'euros, c'est la première ministre qui l'a annoncé, ce qui va leur permettre d'investir sur ce sujet-là, si on relève le plafond de la taxe affectée, il y a plus de 20 millions d'euros qui aujourd'hui écrêter pour l'État, soit ça va augmenter la fiscalité sur l'eau et je crois que c'est ce que personne ne souhaite qu'on touche les consommateurs soit ça va prendre des fractions de taxe affectée à d'autres organismes, l'ouest des par exemple, il y en a d'autres qui aujourd'hui en bénéficient donc on on veut la même chose, je pense que la solution que la première ministre a annoncé et plus efficace pour parvenir à ce que vous recherchez donc toujours avis défavorable. Bien, je crois que tous les arguments ont été données après la rectification de l'amendement de Monsieur Pointereau les trois amendements deviennent identiques, donc je les soumets en même temps on voit donc qui est, pour l'adoption de ces amendements.

les chambres d'agriculture ont signé en novembre 2021, un contrat d'objectifs et de performance avec l'État afin de continuer à porter les politiques publiques du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, or le coût généré par les nouvelles missions du service public confiée au réseau et le surcoût lié à la à sa professionnalisation le réseau fait face aujourd'hui à la hausse de l'inflation, qui met en cause sa soutenabilité budgétaire en ce sens, la hausse du point des chambres d'agriculture de de 75 % décidée le 29 juin 2022 en commission nationale paritaire présidée par le ministère de l'Agriculture entraîne un n'aime pas qu'en année pleine de 11 millions d'euros pour l'ensemble du réseau j'insisterai ici sous la nécessité de contrer l'appauvrissement des chambres d'agriculture, qui n'est pas tenable dans la durée, compte tenu des nouvelles missions majeures que l'État leur a confié, il s'agit d'acteurs locaux essentiels pour les politiques locales de l'État et de nous, qui ne peut pas laisser péricliter le présent amendement vise donc à augmenter les crédits des chambres d'agriculture, de 292 millions d'euros à 303 millions d'euros, soit une hausse de 11 millions d'euros correspondant à l'impact annuel de la hausse de la valeur du point des chambres d'agriculture de de 75 %, cela correspond à un taux de prélèvement de 12 % de la DA TF, soit un taux inférieur à celui de 2015, 2016 et 2017 cette hausse permettra d'aligner les engagements, les objectifs du contrat d'objectifs et de performance avait les capacités financières des chambres d'agriculture, je vous remercie. Merci l'amendement 12 41 c'est qui le présente Madame l'Létard monsieur Delcros, Madame Létard il est défendu. Il est identique en faveur des chambres d'agriculture et donc il est défendu. Défendu l'amendement suivant Monsieur kaput. Oui, c'est moi qui le défend, c'est le même le même amendement que mon collègue Jean-Claude Lenglart hé bien évidement nous nous défendons, compte tenu de l'importance sur le territoires ruraux, des chambres d'agriculture en matière de performances agricoles et de performance aussi écologique. Monsieur Rambo pour le suivant, défendu. Et enfin Monsieur Gremillet défendu monsieur le rapporteur. quelles que soient les chambres consulaires, le problème demeure dans le passé, comme pour l'avenir, s'agissant des chambres d'agriculture, au nombre de 102 donc je rappelle qu'elles sont financées à hauteur de près de 40 par la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, moi j'entends les les arguments puisqu'il émane de tous les bancs, je veux donner quelques éléments, sachant que, effectivement, c'est les, les, les moyens supplémentaires sont demandées par rapport au contrat d'objectifs et de performance tout d'abord, effectivement, c'est l'objet de cet article d'avoir modifié le mécanisme de financement pour se conformer aux objectifs du nouveau code qui a été signé en 2021 et donc 2ème élément, il est prévu une clause de revoyure spécifique en 2023, c'est-à-dire à mi-chemin de la durée de vie du Kopp lequel stabilise le montant de la part de cette taxe versée aux chambres. Je propose donc d'attendre le, comment dirais-je, la clause de revoyure en 2023, d'où la demande de retrait. Monsieur le Ministre, même avis de monsieur le ministre. Donc est-ce que les amendements sont maintenues après la demande de retrait. Dans son. Monsieur. Mais je retire.

Oui, monsieur le président je je vais le retirer aussi. Mais je ne peux pas leur tirer quand même Monsieur le Ministre, que vous entendiez ceci : vous ne pouvez pas demander aux paysans. Devant le défi alimentaire de souveraineté, de sécurité, je vous rappelle que la ferme France tous les ans est en diminution de capacité nourrir nos compatriotes 1er point 2ème point quand on voit qu'aujourd'hui, taxe sur le casse d'art payer 100 % par les agriculteurs 100 pour pour les agriculteurs que vous enlever des moyens de de recherche d'accompagnement des territoires et notamment des chambres d'écriture par rapport aux défis, il y a quelque chose qui va pas, je retire cet amendement mais il est absolument monsieur le Ministre nécessaire de revenir sur le problème du CASDAR de l'argent, des paysans, c'est comme l'eau et du revenir au paysan pour nous hein les enjeux devant nous. Bien, merci les amendements sont donc retirés, nous passons, ensuite à l'amendement 1700 0 17 05 présenté par le gouvernement. Oui, merci Monsieur le Président, très rapidement, c'est un amendement de coordination pour actualiser l'article 15 qui présente les taxes affectées notamment suite à une disposition que nous avons adoptée dans le PLF sur

vise à supprimer le plafonnement qui a été créé par l'intégration de des contributions au de la loi de 2011 pour un montant de 61400 euros en effet, ce principe de ce plafonnement est pour le moins surprenant compte tenu de la situation financière de France compétences de plus le montant de 61,4 millions d'euros et atteint et très éloigné du montant de l'actuel collecte au titre de la formation professionnelle des travailleurs non salariés qui avoisine les 130 millions d'euros, les seules contributions acquittées par les artisans s'élevant elle déjà à 62 millions d'euros, donc, cet amendement vise à supprimer ce plafonnement. défendu, donc avis de monsieur le rapporteur, sur ces trois amendements. Un avis favorable sur la coordination de l'article de l'amendement présenté par le gouvernement, ce qui me permet de dire que les 2 amendements qui sont, qui ont été défendues derrière sont de ce fait largement satisfait.

retiré donc. Nous votons sur l'amendement présenté par le gouvernement, l'amendement 17 05, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. L'amendement 854 monsieur beaucoup. Hé oui, merci Monsieur le Président, le le produit de la taxe sur les transactions financières devrait atteindre l'an prochain de 24 milliards d'euros, ce qui serait un record cette taxe fut créé à l'origine pour participer à la solidarité internationale et réguler modestement quelque peu à la marge la finance mondiale en 2019, la part des recettes de la TTF au fonds de solidarité pour le développement, plafonne à 528 millions d'euros. Or, depuis les recettes de cette taxe ont battu des records en augmentant de plus de 50 % entre 2000 19 et aujourd'hui toute cette hausse au lieu de bénéficier à une politique de solidarité internationale bénéficie au budget général de l'État et au remboursement de la dette donc renforcer cette taxe sur les transactions financières serait un signal fort pour nos partenaires et dégagerait des rendements sans provoquer d'impact négatif sur l'économie française.

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Ensuite 5 amendements qui font l'objet d'une discussion commune, on commence par 2 amendements identiques Monsieur Bonhomme présente le 1er. Oui, monsieur le président, moi c'était un amendement qui a une erreur de de d'ordre parce que il visait à supprimer donc le plafond, mordant mais après ce qui a été dit, je pense qu'il n'a plus de d'être.

par rapport au débat mais cité quand même Jean Launay qui de suit depuis ses de nombreuses années ces ces questions et qui parlait d'une sanctuarisation sinon d'une d'une sacralisation du budget de l'eau. est il est retiré de fait quoi, et c'est la même chose pour le suivant, Monsieur Bockel 923 parce il était identique à celui-là. Oui, retiré OK. Donc ces deux amendements sont retirés, donc on passe à la discussion des suivant Monsieur

Je pense qu'il y a aussi une erreur d'ordre, il s'agissait d'un amendement qui prévoyait un moratoire de 3 ans, par rapport à discussion de précédents sur le plafond mordant, donc il n'a plus lieu d'être, il est retirer. Donc c'est même avis sur les trois amendements, Monsieur le Ministre. Défavorable, donc Monsieur dessus, vous mentez l'amendement ou le retirez retirez monsieur Cozic retirer et Monsieur Bonhomme retirer : il a retiré bien. Nous continuons, nous avons donc ensuite trois amendements, le 841 monsieur Savoldelli. Oui, merci Monsieur le Président. On sait tout ce qu'on est dans un contexte sanitaire qui est inquiétant, du fait de la dans sédentarisation ou en près de 50 ans, les jeunes de 9 à 16 ans aurait perdu 25 % de leur capacité physique, il est grand temps de se donner des moyens pour permettre à toutes et à tous d'accéder à une discipline sportive et de s'y épanouir, cet amendement répond à cette urgence et entend donner les moyens nécessaires pour un réinvestissement massif dans notre politique sportive en s'appuyant sur les leviers fiscaux à notre disposition, en effet, tout le monde le sait ici, où il a été abaissé le plafond de la taxe Buffet afin de tenir compte de la diminution de son rendement provisionnel, ce sont près de 14 4 millions d'euros en provenant de la dotation du programme Sport qui sont venus les les compenser, il apparaît donc pour notre groupe nécessaire d'augmenter le plafond des 2 autres taxes affectées au sport, à savoir, on en parlait tout à l'heure, les paris sportifs et ce hors Paris sportifs dépendant de la Française des Jeux, je rappelle que le plafonnement pour les Jeux, or Paris sportifs et de 71 millions d'euros, alors que le rendement de cette taxe est prévue en 2023 à 246 millions d'euros, nous avons donc une marge considérable en la matière pour les paris sportifs, notre marge de manoeuvre est encore plus large, puisque sur les 180 7 millions d'euros qu'il rapporte chaque année, seulement 34 millions d'euros reviennent au financement du sport, soit à peine 19 % du rendement total en l'espèce, la part de cette taxe accordée au budget du sport reste bloqué à 34 millions d'euros depuis 2018, donc notre amendement demande de manière responsable déplafonnement de 2 des 3 taxe qui ceux qui sont affectés à l'Agence nationale du sport.

donc il s'agit là vraiment du financement de la politique sportive de notre pays à travers la NS qui, vraiment, l'opérateur de la politique sportive dans le pays, je rappellerai simplement que en ce qui concerne le prélèvement de ses 3 taxe il y a simplement 4 ans, les 2 tiers de ces recettes bénéficier aux sports et simplement un tiers tomber dans les caisses de l'État et qui est aujourd'hui la proportion est totalement inversée ces 2 tiers pour Bercy et seul un tiers pour la politique sportive, ce qui veut dire que plus les années passent et puis on s'éloigne du fameux principe le sport finance le sport et en ce qui concerne les paris sportifs en ligne parce que c'est là où effectivement, on assiste à une explosion des recettes cette explosion, c'est plus de 100 % en 5 ans et c'est plus 44 % en 2021 par rapport à l'année 2020 et je rappelle enfin que la NS concerne aussi bien le Paris le le sport de haut niveau que le sport pour tous, et que là on est en train d'aborder le budget de l'exercice 2023 année pré-olympique. Merci, il y a un sous-amendement à cet amendement, présenté par Madame Lavarde. Oui, c'était un moment de de Michel Savin, dont nous connaissons l'expertise en matière de sport qui vise en fait à à, enfin, poursuit le même esprit que celui défendu à l'instant par monsieur Lozach mais tout en étant quand même beaucoup plus raisonnable, puisque là il limite le prélèvement à hauteur de 14 4 millions d'euros, et c'est un montant qui en fait équivalents à l'effort que l'État et a dû faire en venant abonder les crédits pour compenser, en fait, la baisse de la taxe Buffet le l'effort de de l'État, et là, c'est-à-dire que moins on maintient, mais il semble oh cosignataires de ces amendements qu'il faut faire plus notamment pour soutenir les équipements de proximité. Merci enfin 4ème amendement monsieur Oui, l'amendement de notre collègue Laurence Harribey, là il s'agit, au contraire, enfin, au contraire, je dirais, en complément, il s'agit d'un déplafonnement des autres Paris qui sont exploités, qui sont gérés par la Française des Jeux et je dirais que ce type de proposition n'a rien d'exceptionnel puisqu'on a connu ça par le passé, notamment pour le financement de la construction et de la rénovation des stades pour la Coupe d'Europe de foot en 2016 il y avait eu à ce moment-là, un prélèvement exceptionnel de 0 3 % sur les jeux de la Française des Jeux en 2011, qui avait été prolongé en 2017 et je dirais que cet amendement, hé bien il est, il peut être destiné en particulier à financer le fonds héritage olympique afin que celui-ci se pérennise véritablement une fois les Jeux olympiques derrière nous. Merci donc sur ces trois amendements et le sous-amendement, monsieur le rapporteur. de enfin, demande de retrait ou avis défavorable, en fait, ces amendements posé la question concrète du financement du sport

c'est plutôt des crédits budgétaires qu'il faut développer non mais autant se dire les choses, il faut qu'on essaie d'être en cohérence dans nos demandes, je note, parce que il faut parfois aussi dire les choses que pour 2023 la subvention qui a versé à l'Agence nationale du sport

je crois que c'est un sujet important, effectivement, vous l'avez dit, nous sommes dans une, dans des années pré-olympique et il faut essayer de faire le lien entre la développement de la pratique du sport, l'encouragement aux pratiques sportives et la mise à niveau des installations sportives parce que c'est utile d'avoir une France qui soit au moins égal dans la pratique des sports dans tous les territoires, comme on le propose, par exemple, et de la même manière, avec une forme de cuménisme même s'il a des freins parfois sur la culture ou d'autres pratiques. Merci monsieur le ministre. moi je veux rappeler que l'Agence nationale du sport, elle est notamment financée par la taxe Buffet qu'il y a cette année une baisse du rendement de la taxe Buffet et que nous faisons plus que compenser cette baisse du rendement de la taxe Buffet par des crédits budgétaires supplémentaires, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'on on transforme une ressource variables incertaine liée à une taxe affectée en ressources, certaines avec des crédits budgétaires et ont fait plus que compenser la baisse. Du rendement de la taxe Buffet 2ème chose je veux rappeler que l'Agence nationale du sport bénéficie d'une enveloppe importante pour les équipements de proximité et qu'elle dispose encore de fonds du plan de relance pour financer aussi ces équipements et donc pour ces raisons avis défavorable. Bien, donc on a un avis défavorable, une demande de retrait ou avis défavorable sur tous ces amendements peut-être avant de passer la parole, je vais demander aux de des amendements si les maintiennent vous le maintenez. Savoldelli, il est maintenu, monsieur Lozach, il est maintenu le sous-amendement. Le sous-amendement est maintenu.

Quand même, je la prends pas souvent, alors attendez. Bien je je ne vais pas prendre les deux minutes, rassurez-vous, j'ai bien entendu les les arguments du du rapporteur Huchon évidemment vaut mieux des crédits affectés mais la problématique de la politique, du sport, elle est très importante, pas seulement parce qu'il y a les Jeux olympiques, la France est pas vraiment un pays sportif pourquoi parce que, pour que nos collectivités se dotent d'équipements. C'est le parcours du combattant, il faut les chercher un peu essai des Ciel parfois de la DETR et quand tu l'la NS et présente, c'est très bien mais c'est rarissime, j'ai entendu parler d'équipements sportifs de proximité, vous allez faire le tour de vos départements pour savoir combien de SP ont pu être financées par la NSA, moi dans mon département et se comptent sur les doigts d'une main, OK, donc plus la NS aura de moyens, mieux ce sera, parce que le sport c'est pas seulement un vecteur de cohésion sociale, c'est un vecteur de bien-être personnel et caetera et caetera, on le sait tous, donc il faut plus de moyens pour le sport, alors ça peut passer évidemment par des crédits affectés, j'ai entendu aussi le ministre, mais les arguments de nos collègues qui ont présenté des amendements pour mieux dotés via la taxe Buffet là NS sont tout à fait acceptable aussi. Bien, merci, donc on va passer au vote sur ce monsieur Lozach. Simplement une réponse à ce que disait Monsieur le Ministre tout à l'heure, bon bien sûr on préférerait des crédits budgétaires à des crédits extrabudgétaires mais quand tout à l'heure, il dit que, effectivement, la faiblesse du produit de la taxe Buffet cette année est compensé par l'État, je voudrais simplement rappeler que les 14 il y a eu 4 millions d'euros qui sont prévues, effectivement, par l'État, c'est un prélèvement sur d'autres actions de la politique sportive du programme 219 donc, ce n'est pas une dotation supplémentaire de l'État, mais un simple prélèvement sur d'autres actions de ce même budget. Bien, donc nous allons passer au vote sur ces amendements, dont l'amendement 841 présenté par Monsieur Savoldelli qui est pour.

Qui s'abstient, il n'est pas adopté et sur le dernier amendement 1029 même vote même vote, ils ne sont pas adoptés donc nous passons au 14 76 madame DeMarco. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis sa création, la contribution à la vie étudiante de Campus est extrêmement contestée par les étudiants dépourvu de progressivité ce barème frappent indistinctement les étudiants, quelles que soient leurs moyens, elle rajoute ainsi de l'injustice fiscale au système d'aides publiques à la vie étudiante, qui nécessite une réforme d'ampleur d'ajournement de la réforme des bourses Chiquita sociaux maintient aujourd'hui un régime qui manque de progressivité et qui rend difficile l'aide aux étudiants de classes moyennes se trouvant juste au-dessus des seuils d'éligibilité, c'est par exemple le cas dispositif exceptionnel de repas un heure qui ne bénéficie qu'aux étudiants boursiers, par ailleurs, l'inflation, contre 1 considérablement les Crous dans leur gestion, avec des répercussions sur la vie sur des étudiants non boursiers, devant la commission de la culture, notre rapporteur d'ailleurs souligné que la non-indexation de la S. P loué au Crous sur le volume de repas fournis étaient anormales, elle stagne aujourd'hui à 300 millions d'euros. La contribution de la vie étudiante du campus, c'est également contesté dans son utilisation et dans sa gestion, l'opacité et l'affectation de la Fed, question de son produit régulièrement pointée du doigt par les étudiants qui dans les faits, ne constate pas d'amélioration des services universitaires, il n'est pas acceptable que l'effort supplémentaire demandé à nos étudiants puissent servir à compenser le désintérêt là si ce monde l'est en la matière, je rajoute dans le cas d'étudiants admis tardivement au bénéfice d'une bourse essayant à acquitter de la CDEC au moment de l'inscription le remboursement relève du parcours du combattant, nous proposons donc dans cet amendement de rétablir l'intégralité des recettes de la CVAE c'est au Crous et aux établissements de l'enseignement supérieur. L'amendement veut donc rétablir le montant initial de la CDEC toutefois le montant qui est inscrit correspond au rendement attendu de la CBC, qui est d'ailleurs payé par les étudiants eux-mêmes et qui est reversée aux établissements et aux Crous. En conséquence, votre amendement revient à vouloir augmenter un montant payé par les étudiants, ce qui me paraît être le contraire de son objet d'une demande de retrait. Merci monsieur le président, j'avais pas prévu forcément de prendre la parole, mais je peux pas laisser dire que la création de cette contribution sur la vie étudiante est venue grever le pouvoir d'achat des étudiants. Parce que quand elle a été créée, c'est parce qu'on a supprimé la taxe sur la sécurité sociale étudiante de 217 euros qui touchait les étudiants pour accéder à la sécurité sociale, on sait en fait objectivement que ça financer autre chose, je vais pas rentrer dans les détails, mais enfin à travers les mutuelles étudiantes, les syndicats étudiants, c'était une taxe pour soi-disant accéder à la sécurité sociale en réalité pour financer plutôt des actions politiques, on a supprimé cette taxe en 2017 on a supprimé la taxe pour accéder à la sécurité sociale et maintenant les étudiants sont affiliés à la Sécurité sociale gratuitement et on a créé cette contribution, qui est de l'Ordre de quatre-vingt-dix euros qui ne touche pas les étudiants boursiers, par ailleurs, qui permet de financer des projets concrets pour la vie étudiante sur les campus en matière de santé en matière de sport et et d'autres projets, donc à la fin, le pouvoir d'achat des étudiants entre ces 2 mesures s'améliore, ils ont moins de taxe à payer et donc pour reprend ce que disait le rapporteur général, on relève le plafond au niveau de ce qu'on collecte en matière de CV E c'est c'est de bonnes pratiques et de bonne gestion des finances publiques que d'avoir un plafond sur les taxes affectées mais évidemment sur la vie étudiante, tout ce qui est payé par les étudiants pour la vie étudiante va à la vie étudiante et chaque année on relève le plafond au niveau du rendement de la contribution, c'est le cas encore cette année, donc avis défavorable. D'un double avis défavorable, je le soumets aux voix qui est pour. Qui est contre. S'abstient, il n'est pas adopté ensuite nous abordons 13 amendements en discussion commune. Les. Nous démarrons par 6 amendements identiques monsieur Arnaud pour le premier, le 621. de 300 points de contact par 2500 élus consulaires et touche un 1000000 800 1000 entreprises artisanales de France, il s'agit simplement de maintenir les moyens de l'année 2022 pour 2023 afin de consolider les efforts faits par ce réseau dans le cadre notamment de la transposition et de la mise en oeuvre de la loi, pacte qui a déjà subi une restructuration très importante, il ne s'agit pas durant l'année 2023 d'affaiblir ce réseau particulièrement utile pour les entreprises de proximité que sont les entreprises artisanales. Merci le 674 Monsieur Ruquier défendu le 741 monsieur qui a pu. Il a été doublement défendu le bus, c'est effectivement de ne pas affaiblir les chambres des métiers de l'artisanat, au moment où elles ont déjà procédé à des mutations importantes à la demande de l'État.

Oui, je suis président, je défends les deux en même temps très rapidement, pour vous dire que les chambres de métiers et de l'artisanat, ont une place et un rôle essentiel pour accompagner les entreprises artisanales qui sont souvent de petites entreprises dans la difficulté actuelle la pandémie puis aujourd'hui la crise de l'énergie, donc il est important que leurs moyens soient préservés, de même que dans le cadre de la réforme de la loi, pacte qui vise à supprimer un certain nombre de formalités administratives, les chambres de métiers, reste un acteur important. on continue avec les amendements qui sont dans cette discussion commune, il y en a 6 autres. 389 allez-y. dans la même veine, afin de préserver les ressources des des CM1 en limitant cette fois, la baisse de la taxe affectée à à cette à 7 millions d'euros en 2023. Monsieur Ruquier défendu monsieur kaput défendu monsieur boulot défendu également je pense monsieur monsieur il est pas soutenu le suivant est monsieur Calvet, l'amendement de repli défendu donc monsieur le rapporteur sur tous ces amendements. je pense j'ai on a parlé des chambres d'agriculture tout à l'heure, on parle là des chambres de métiers, ce qui me paraît aujourd'hui indispensable, c'est que ce qui est dans la trajectoire de des dispositions qui étaient prévues et des dispositifs d'évolution des trajectoires de financement ou du concours de l'État aux chambres de métiers doit être, comment dirais-je, régler avec entre l'État et les chambres de métiers, une fois que ce sera définitivement scellé, c'est plus facile pour le Parlement de confirmer ces éléments et je dis une 2ème chose, on voit la difficulté finalement des orientations qui vise à réduire les moyens, je prends un exemple comme ça, vous verrez les chambres de métiers, de devoir de commerce devait voir là aussi avec la loi pacte les moyens diminuer ça a commencé à diminuer et lorsqu'est arrivée la crise sanitaire pour le plan de relance, vous vous êtes tout de suite, appuyé sur les réseaux des chambres de commerce et vous avez vous-même reconnu que heureusement qu'elles étaient là, voilà, donc c'est finalement il faut être attentif aux dispositifs et essayer de trouver le bon équilibre, c'est ce à quoi nous vous invitons si tout le monde suit l'vie avec un avis favorable. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, les chambres des métiers de l'artisanat, elle joue un rôle essentiel dans notre pays, vous me permettrez de saluer toutes celles et tous ceux qui les font vivre il y a une trajectoire d'ici à 2027 effectivement de baisse du plafond de la taxe qui leur est affecté, mais c'est parce qu'il y a dans le même temps, des dépenses en moins pour les CM1. Pour 2 raisons : 1 parce qu'il y a eu une réorganisation du réseau et je rappelle qu'on est passé de quatre-vingt-trois entité coordonné par une assemblée des chambres, un réseau de dix-huit chambres régionales et de 2 chambres locales coordonné par CMA, France 2 il y a eu des évolutions en matière de mutualisation et de. Gouvernance ça va avec, donc ça c'est pour le volet rationalisation économique et ensuite il y a eu la loi pacte qui a transféré un certain nombre de compétences des CMA on a transféré les Centres de formation et d'apprentissage aux branches, on a transféré l'enregistrement des contrats d'apprentissage aux opérateurs de compétences et on a substitué les registres dématérialisée au centre de formalités des compétences, donc il y a eu une réforme avec la loi, pacte qui fait qu'on a transféré des compétences des CMA à d'autres opérateurs, il y a eu un effort et je veux le saluer de réorganisation de mutualisation et d'économie, ce qui fait que tout ça a fait baisser les charges, il est le besoin de dépenses des CMA et donc, en face, on baisse le plafond de la taxe affectée mais le plafond, la baisse de ce plafond de taxe affectée correspond à une baisse de besoin de financement pour les CM1, il y a pas de fragilisation du réseau c'est équivalent, donc moi je veux vraiment le rappeler, on a souvent ces débats ici on appelle à des économies des réorganisations des modernisations, des mutualisations pour améliorer la trajectoire des finances publiques là en l'occurrence il y a un gros effort qui a été fait et encore une fois le la baisse du du plafond de la taxe affectée correspond à cet effort, donc il n'y a pas lieu de le relever, ou de le supprimer ou de supprimer la trajectoire qui a été acté, donc avis défavorable. Monsieur Gremillet. Oui, mais monsieur le président, Monsieur le Ministre Monsieur rapporteur général, chers collègues, moi je me réjouis la position notre rapporteur général, monsieur le Ministre. Les choses ont changé : aujourd'hui, il y a un défi, le défi, c'est de repositionner de reproduire dans nos territoires, ce qu'on a pu été capable de produire et au moment où il y a besoin d'injecter de soutenir des initiatives, on supprime les moyens c'est pas cohérent, donc effectivement, Monsieur le Ministre, entre ceux qui vous avez décidé, dans un autre temps le le monde a changé il y a une stratégie politique, y compris du gouvernement, y compris de l'Europe et vous êtes à l'inverse de ce que vous décidez, au niveau de l'accompagnement des chambres de métiers, moi je soutiens vraiment ces amendements, je remercie le positionnement favorable de notre rapporteur général merci. Monsieur le Président, simplement pour dire que si la régionalisation entraîné effectivement des économique hein, mais lundi dans le Ministre, ça se saurait, on l'a bien vu avec le regroupement des régions de France, ça n'a entraîné absolument connaît économie, par contre, ce que nous souhaitons, Monsieur le Président, c'est que les chambres de métiers de l'artisanat reste extrêmement extrêmement présente sur le territoire, 1er élément 2ème élément sur la dématérialisation des formalités administratives oui c'est en cours mais mais la validation de l'ensemble des inscriptions doit se faire toujours par des chambres de métiers, ce n'est pas lié, pays qui le fait donc ça veut dire que les chambres des métiers ont encore un rôle important. donc, nous allons passer au vote sur les 6 amendements. Les six premiers identique, 621 674 741 859 933 et 1411 et 1411 avec un avis favorable de monsieur le rapporteur et défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés donc les suivants tombe, je mets aux voix, l'article 15 qui est pour l'article 15, ainsi amendé. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté après l'article 15. Nous démarrons avec 2 amendements en discussion commune le 1500 Monsieur Cosic Monsieur Féraud Monsieur Covic. Oui, merci Monsieur le Président, donc cet amendement propose l'extension de la redevance pollutions diffuses qui aujourd'hui ne couvre que le volet phytosanitaire, il s'agit donc d'aller plus loin dans la lutte contre les micro-polluants qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années, comme les dernières études sur la qualité de l'eau, le démontre. Grâce à cette amendement cette extension de la redevance sur les donc appliquer au metteur sur le marché, produisant, vendant ou important des produits contenant un ou plusieurs polluants à à compter du 1er janvier 2023. Des produits comme certains médicaments biocides. Ménage même ménagers produits comestibles cosmétiques ou d'hygiène seraient concernées en appliquant un taux modulée selon la nocivité de la de la substance indésirable et cumulable selon le nombre de substances cette redevance permettrait, donner un signal prix qui incite à l'éco-conception par les industriels et de mobiliser de nouveaux financements collecté par les agences de l'eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics, de gestion de l'eau sur l'ensemble du territoire national,

Et est défendu, avis de monsieur le rapporteur défavorable, monsieur le Ministre défavorable, donc un double avis défavorable, il est maintenu. Donc je le soumets au au voile le 1572 qui est pour.

il y a un amendement identique, excusez-moi monsieur Gremillet. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre ne sera rapporteur général, chers collègues, cet amendement c'est un amendement de ça c'est planification qui consiste tout simplement à ne plus verser d'acompte sur la taxe de redevance mais que, effectivement, ce soit payer une seule fois c'est ça n'a aucun impact budgétaire, c'est une mesure de simple simplification. Merci monsieur le président, je ne peux qu'être défavorable à cet amendement, après vous avoir longuement écouté sur les agences de l'eau, ce que ça viendrait fragiliser les agences de l'eau. Ce que la compte lors et aujourd'hui versé. Donc, sauf si vous avez été convaincu par mon argument sur le fait que le fond Vert permettra de soutenir les agences de l'eau et du coup il y a moins besoin de moyens, mais sinon, je ne peux pas être favorable à cet amendement qui avis défavorable. Monsieur le rapporteur.

à développer l'argument parce que là où la ficelle est un peu trop grosse, compte tenu des moyens que vous enlever tous les ans aux agences de l'eau, mais on n'a pas le temps, j'ai entendu le président je me tais, je leur dire.

liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour, en fait, ça vise tout simplement à concrétiser une recommandation du défenseur du droit qui a été formulée en 2014 qui l'a réitéré en 2016 puisque cet axe cette exonération s'applique mais au coup seulement aux conjoints étrangers de ressortissants européens qui résident en France, le défenseur des droits considère à juste titre, que cette différence de traitement constitue une discrimination à rebours fondée sur la nationalité est prohibé par le droit européen d'ailleurs notre assemblée avait adopté une disposition similaire à cet amendement en 2021, mais qui n'avait pas été reprise par l'Assemblée nationale. Merci, monsieur le rapporteur. Demande de retrait. Demande de retrait. Le ministre même avis donc. Une double demande le retrait, il est maintenu, je le soumets aux voix. Qui est favorable à cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Amendements suivant 3 amendements en discussion commune le 77 Monsieur Non, cette lecture simple je pense monsieur le président, mais on nous reproche souvent, monsieur le président de d'engager trop de dépenses, ici, il vous est proposé de réaliser des économies en supprimant une niche fiscale relative la taxation à l'imposition des indemnités de rupture conventionnelle, il y a pas de raison que comme les autres revenus des salariés ne soient pas imposable.

Monsieur le Président, cet amendement prévoit d'appliquer aux indemnités de rupture conventionnelle qui sont versés aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat, qui sont des agents publics, en vertu d'une jurisprudence constate du Conseil d'État, le même régime fiscal qui est prévu à l'article 80 du des sièges du code général des impôts, en effet, tous les agents publics et salariés relevant du droit du travail bénéficie d'une indemnité de rupture conventionnelle exonérés dans la limite d'un plafond, sauf les directeurs généraux d'office public de l'habitat, il ressort clairement des débats parlementaires qui avait lieu au moment de la loi Macron que le législateur n'a pas entendu traiter différemment les directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie des directeurs généraux d'office public de l'habitat, pour ce qui concerne le régime de l'indemnité de rupture

de l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle, cela constitue, me semble-t-il une exception injustifiée au regard de la généralisation de l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle et cela crée surtout une rupture d'égalité devant la loi fiscale et les charges publiques. Une demande de retrait sur le 77 qui créerait, comment dirais-je à un dispositif que je qualifierais de bancale par rapport à l'exonération, notamment lorsqu'il y a licenciements puisque c'est prévu un avis favorable pour l'amendement 1692 puisqu'il n'y a, de notre point de vue, effectivement, de mon point de vue, pas de raison d'avoir un traitement différencié selon les personnels, des chambres consulaires je vais demander au gouvernement son avis sur le mille sur le 224 pardon parce qu'il est effectivement assez difficile à comprendre les raisons d'un traitement différencié pour ne pas dire obscur quand si obscur, j'ai aussi besoin d'avoir les lumières du gouvernement. Monsieur le Ministre. Il peut y avoir des raisons de douter de de l'intérêt de cette exonération qui est par ailleurs coûteuse pour les finances publiques de 145 millions d'euros, le l'amendement de Monsieur Calvez proposent de la supprimer mais je crois que cette réforme, si elle venait à être mise en place doit être concertée quand même avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble des acteurs concernés et ne je ne suis je ne pense pas souhaitable de supprimer cette exonération des aujourd'hui, mais ça peut faire partie des sujets et je pense que ça fera partie des sujets sur lesquels nous serons amenés à travailler dans l'attente, le traitement différencié des CMA, donc ça c'est le l'amendement qui a été défendu par Monsieur Rambo, je donne un avis favorable à cet amendement il y a une situation particulière, on en a parlé tout à l'heure dans les presser dans un moment de restructuration des CMA qui justifie cette ce traitement différencié, en revanche, on ne peut pas dire qu'il y ait le même besoin pour les directeurs des OPH puisqu'on n'est pas dans la même situation que les CM1, il y a pas les mêmes Restructuration aujourd'hui, s'agissant des OPH que pour les CMA donc je donnerai un avis défavorable à l'amendement de Madame Estrosi Sassone pour ces raisons. Bien, monsieur le président de la ou de la parole. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi, moi je j'interviens pour pour soutenir l'amendement de Michel Canevet, du groupe d'union centriste, je pense que quand il s'agit d'indemnités conventionnelles d'une rupture conventionnelle, les indemnités pour moi en tout cas moi je suis favorable à ce que tous les revenus soient imposables et donc quand on touche une année petit conventionnelle qu'on a décidé de se se mettent d'accord avec son employeur pour quitter, je ne vois pas pourquoi on exonère c'est revenu d'impôt, on cherche des recettes, hein, ce ministre une petite jours est-ce que vous avez des recettes, hop là en l'occurrence, on en a une, je ne vois pas pourquoi on ne voteraient pas cette exonération, en tout cas pour ma part, je la soutiens. Bien, donc on va passer au vote sur ces amendements, donc le 1er le 77 avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté ensuite le 16 192 avec un double avis favorable qui pour. qui est contre. Qui s'abstient. Pas adopté le 224 donc un avis défavorable du gouvernement et la commission. Même avis. Donc, il est pour cette il est maintenu, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Pour le seize 92 Monsieur le Ministre, vous devez lever le gage. Vous vous levez le gage bien. sont ensuite 5 amendements en discussion commune. Donc, nous commençons avec le 821 monsieur Bouquet. Oui, merci Monsieur le Président, très rapidement, cet amendement, qui propose le doublement de la taxe sur les transactions financières qu'on a évoqué tout à l'heure et l'intégration des transactions intra-journalières, selon le jargon en usage la spéculation va bon train selon tous les spécialistes, on le constate régulièrement et je rappelle que l'augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières fut une proposition remise au goût du jour avec la Convention citoyenne dont on sait quel sort lui fut réservé.

puisque le le premier bien sûr concerne la la hausse du taux de la taxe sur les transactions financières, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, et compte tenu des des profits records et des dividendes distribués cet amendement propose donc de de rehausser le taux de taxation des transactions financières de 0 3 % à 0 5 % et le le second amendement qui complète le premier propose d'élargir le Champ, donc de la taxe sur les transactions financières aux transactions dites infra-infrajournalières qui inclurait ainsi les transactions intervenant avant le transfert de propriété à l'acquéreur, ce qui, je le rappelle, avait été votée par le Parlement en 2016, je vous remercie. Oui, c'est aussi énormément, qui propose d'augmenter la taxe aux transactions financières à 0 5 % nous avons toutes et tous pu constater l'impact de la pandémie sur le système de santé mais si le système, le système de santé français a souffert et souffre encore l'impact dans certaines parties du monde a été catastrophique, la pandémie a déstabilisé la lutte contre les maladies évitables, je parle du VIH de la tuberculose ou du paludisme, entraînant un risque élevé de reprise de ces épidémies, l'extrême pauvreté a progressé dans le monde, pour la première fois depuis les années 90 et l'atteinte des objectifs de développement durable et plus que jamais compromise à 8 ans de l'échéance de l'Agenda 2030 l'augmentation que nous proposons de faire passer avec l'augmentation que nous proposons le rendement, la taxe passera à 3 7 milliards d'euros, contre deux deux actuellement, cela représenterait 5 milliards d'euros supplémentaires pour la politique de développement française pour renforcer les financements allant au fonds de solidarité pour le développement pour principalement financé les dons vers les priorités fixées par la France que sont notamment la santé, le climat et l'éducation qui bénéficie au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme à United au fond Vert pour le climat au partenariat mondial pour l'éducation, ces institutions beaucoup sédation beaucoup se consacre à rattraper le retard dû au Covid et se mobilisent dans le renforcement des systèmes de santé afin de préparer la communauté internationale aux prochaines pandémies l'amendement suivant a déjà été défendu mais c'est aussi pour intégrer les transactions intra-journalières à l'assiette de la taxe sur les transactions financières, c'est-à-dire autres actions intervenant avant le transfert de propriété à l'acquéreur, on a donc 2 objectifs : avec cette amendement augmenter les recettes de la taxe, outil de justice fixe à 2 fiscal au soutien large et transpartisan et se conformer à l'objet 1er de l'instauration de la taxe, en luttant contre la spéculation boursière en l'état la taxe les transactions financières n'atteint pas efficacement ce second but, je vous remercie.

je ai soumet au vote donc le 820 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 481 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté le 530 même vote même vote le 563 même vote. Et le 482 même vote. Même botte. Donc, ensuite, nous passons à l'amendement 1282 Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le le président c'est un amendement pour faire de suppression d'une exonération pour faire participer le fret maritime à hauteur de son impact environnemental, le régime fiscal applicable aux activités navigation maritime au transport de marchandises sur ces voies, questionne la pertinence de la politique environnementale française responsable une pollution dans l'impact environnemental est supérieur à celui de l'automobile, le transport maritime demeure toutefois bénéficiaire d'une exonération de taxe sur les carburants, alors que l'acheminement de marchandises se fait essentiellement au moyen du fret maritime, les émissions d'oxyde de soufre qui génère et leurs lourdes conséquences sanitaires, écologiques, ne peuvent que contrasté avec la faiblesse des réglementations sur ces carburants afin, du coup, de rétablir une cohérence dans le traitement de l'urgence environnementale par la France le présent amendement propose que le fret maritime, participe à la hauteur de son impact sur les écosystèmes à l'effort fiscal français en faveur d'appréhension écologique en ce sens, il est estimé nécessaire que ce secteur soit concerné par les prélèvements de taxes sur les carburants, alors que les armateurs français au 1er rang desquels CMA-CGM réalisent des profits records 18 milliards pour mémoire de dollars pour en 2021, le maintien de cette exonération paraît d'autant plus aberrant merci. Un avis défavorable, Monsieur le Ministre, défavorable, donc un double avis défavorable, je le soumets aux voix qui est pour.

trouver un moyen de, de, de financement, notamment de la fille de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, aussi appelé également taxe d'aménagement du territoire et du par les concessionnaires d'autoroutes a raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers, elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers sur les péages perçus, mais effectivement, quel que soit le type des véhicules et quelle que soit l'impact de ce véhicule justement sur le le l'usure je dirais de de des des routes le présent amendement propose pour les poids lourds, notamment de plus de 7 5 tonnes un montant de taxe avec un coefficient multiplicateur de trois par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules, une telle mesure permettra de faire contribuer l'ensemble des poids lourds, y compris notamment les pavillons étrangers à l'amélioration des infrastructures de transport, en accroissant les moyens de la FIT, cette proposition est inspiré d'une proposition de France Nature Environnement, merci. Alors un avis défavorable je mais je, je vais dire que toute modification finalement de la fiscalité, notamment la fiscalité qui est spécifique aux sociétés gère d'autoroute entraîne et vous le savez, sur le fondement de l'article 32 des contrats de concession, un droit à compensation susceptible et là c'est on rentre dans les négociations. à risque et, notamment, le risque c'est de d'avoir un impact en rebond sur la hausse des tarifs de péage et je pense que l'esprit de votre amendement, c'est plutôt l'inverse, et j'ai entendu à une certaine époque, une ministre, être très volontariste et très allante pour faire plier les sociétés d'autoroutes, enfin le pensait-elle et à l'époque, le droit des contrats, il est assez difficile à modifier, parce que c'est un accord entre les parties, donc avis défavorable. Monsieur le Ministre, même avis du ministre. Le second. j'ai rapidement, j'entends ce que dit le le rapporteur, effectivement, ça pose réellement la question des des concessions autoroutières et ça me permet d'ailleurs de de rappeler, en tout cas de demander au au Ministre justement ces intentions par rapport à ces concessions, dont on sait que certaines arrive à échéance et dont d'autres arrivent à échéance, donc assez assez rapidement et donc à un moment donné, il faudra quand même avoir une vraie décision et un vrai questionnement sur la question de ces concessions, puisqu'on voit bien que on est totalement pieds et mains liés par rapport aux possibilités qu'on peut avoir à faire et notamment sur les questions à la fois de taxation et de et de manière dont on peut intervenir sur ces concessions. Monsieur Gontard donc l'amendement est maintenu. Oui, donc je le soumets aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Amendement 1281 Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président, de nombreuses compagnies aériennes effectuent des vols à vide ou très peu rempli, faute de passagers et contraints par la réglementation européenne sur la conservation des slots créneaux horaires qui autorise une compagnie a décollé d'un aéroport où il a été rire à un moment précis, si la réglementation européenne oblige pas réellement la compagnie à opérer des vols à vide, elle l'empêche d'annuler massivement des vols insuffisamment remplis pour être profitable, or un vol insuffisamment remplis pour être profitable, est un vol quasiment vide, pour sûr rempli à moins 30 % 30 % de sa capacité maximale, le droit français, à l'air que droit aux Européens, les vols à vide sont une aberration écologique, on le sait tous, on a plein d'exemples, à laquelle il faut évidemment mettre un terme dans les plus belles c'est ce pourquoi nous proposons cette mesure pour mémoire un avion émet 9 kilos de CO2 par 100 kilomètres par passager en moyenne ainsi un vol à vide intra- européen, par exemple, un Paris Athènes qui aurait pu accueillir 236 passagers produit 45 tonnes de CO2, cet amendement a donc pour objet d'instaurer une taxe sur les sièges sans passagers dans les avions pendant le pendant de la taxe sur les billets d'avion alors a pour double effet de limiter les vols en sous-effectif, qui coûte cher, écologiquement et économiquement notamment carburant mais aussi de forcer les compagnies aériennes à mettre en vend des billets moins chers pour favoriser le remplissage de leurs avions et cette mesure prend donc un double effet à la fois un intérêt écologique mais aussi un intérêt social permettant compatriotes les plus modestes de voyager à des prix abordables merci. Merci, monsieur le rapporteur. Demande de retrait. Demande de retrait. Le ministre même même avis. Vous mettez l'amendement président Gontard, donc je le sommet on voit qui est pour.

Monsieur le Ministre, cet amendement est présenté au nom de la commission de l'aménagement du territoire, il a été voté à l'unanimité, il vise à sécuriser les ressources de l'Agence de financement des infrastructures en France la fuite l'Agence concourent au financement des projets d'infrastructures de transport, d'ampleur, vous le savez, qui ont pour caractéristique de s'inscrire dans le temps long, pourtant la fille bénéficie de ressources qui sont pour plusieurs d'entre elles, incertaine, à l'image de la contribution du secteur aérien, ou bien des amendes radars radars dont elle est la dernière bénéficiaire, une fois que les répartitions sont faites, c'est pourquoi, alors que la décarbonation du secteur des transports est une priorité, il est important de sécuriser ses recettes, c'est pourquoi le présent amendement propose, dans le cas où certaines recettes viendrait à manquer, je dis bien dans le cas où certaines recettes viendrait à manquer d'affecter davantage de TICPE à la fuite afin de lui permettre de respecter sa trajectoire de dépenses, je voudrais préciser, et sans doute à à monsieur le rapporteur général que bien sûr nous avons auditer la fuite et nous avons bien noté que, il y a des crédits aujourd'hui qui sont disponible mais tous les crédits en fait, ils sont bien bien gagés mais ne sont pas forcément engagée et c'est toute la différence, ça veut dire qu'il y a une difficulté à mettre en oeuvre les conventions et à mettre en oeuvre les véritables programmes qui nécessite effectivement ces financements il y a une lourdeur aujourd'hui juridique et qui met en difficulté également l'Afrique mais ça n'a rien à voir avec les montants et les dépenses qui sont, qui doivent être alignés par rapport à à ces programmes là, c'est pour ça qu'il faut vraiment sécurisé la trajectoire et les ressources financières de la

parce qu'effectivement la situation de la fuite, il y a encore quelques années, chaque PLFR de fin d'exercice, il fallait jouer un peu aux sauveteurs dans ce PLF, les choses se sont améliorées, mais j'ai bien compris que c'est, c'était le sens aussi de votre propos, si on regarde cette année, ça doit quand même être portés à notre connaissance, la fuite a dû annuler en fin d'année des montants très significatifs de crédit lors du 4ème budget rectificatif pas parce qu'elle manque de recettes, mais au contraire parce qu'elle n'est pas en mesure de consommer ces crédits et en 2022 par rapport aux prévisions du budget initial Lafitte aura annulé 500 millions d'autorisations d'engagement et 260 millions de crédits de paiement. Ce qui me paraît raisonnable et équilibré, c'est avant de s'engager dans une procédure qu'on pourrait appeler de sécurisation des recettes en 2023 de l'agence, voyons si et comment elle procédera effectivement aux dépenses dont elle dispose et me semble-t-il, il sera où il serait temps ensuite dans un PLFR d'apporter la le le le le les modifications nécessaires et de rectifier la trajectoire, raison pour laquelle j'aurais un avis de retrait. Monsieur le Ministre. Même avis du ministre Monsieur Gillet. Retrait. Donc, l'amendement est retiré, donc nous passons à l'examen de l'article 16, j'ai une demande de prise de parole de Madame Jasmin. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, là si votre attention sur les mesures que vous envisagez de prendre qui priveront de 300 millions d'euros les fonds nationaux d'aide à la Pierre, un quart de la collecte de la participation des entreprises à l'effort de construction, c'est le budget des programmes ANRU Action coeur de ville, plan d'investissement volontaire pour les départements d'outre-mer et les régions d'outre-mer, hé bien qu'il se rende très fortement ce sera quand même la catastrophe, il est urgent de prendre en compte les situations qui sont clairement identifiées et les besoins, je crois, Monsieur le Ministre, que vous devez au contraire abondé de 150 millions d'euros. Ces fonds nationaux d'aide à la Pierre pour permettre que l'ensemble des mesures qui sont prévues soient réalisables et réalisées, je vous remercie. Merci madame Jasmin, donc nous avons 2 amendements en discussion commune présentée par Madame Létard par la présidente l'État. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, monsieur le rapporteur général, chers collègues, cet amendement a pour vocation de corriger dans ce PLF une incongruité aux effets dévastateurs concernant un acteur central du logement social en France, le logement 1er poste de dépenses des Français, des foyers français n'est-il pas l'une des priorités du gouvernement, mettre à leur disposition des logements abordables n'est-il pas l'une des clés pour améliorer le sort des salariés aux revenus modestes de notre pays et à nos travailleurs clés dans les territoires en tension à à l'heure où plus de de 2 millions de foyers sont en attente de logements sociaux, le soutien de salariés et leur pouvoir d'achat sous l'influence de l'inflation est au centre de nos préoccupations, il paraît dangereux de vouloir déstabiliser ce modèle vertueux du développement du logement social, en effet, Action logement est aujourd'hui un producteur essentiel de logements sociaux sur les 5 dernières années, c'est plus de 500000 logements construits 400000 ménages logés 800000 garantit le locative Visale accordé, et j'en passe, or depuis 2020 Action Logement service a connu plusieurs prélèvements exceptionnels, je souligne ici l'emploi de guillemets dont 1,5 milliard au profit du Fonds national des aides au logement, ce qui a conduit à mobiliser intégralement le surplus de trésorerie d'ALS auquel vient s'ajouter la prise en charge par Action logement d'une partie des contributions versées à la CG 2 Alès par les bailleurs sociaux afin de financer le Fonds national d'aide à la Pierre, pour un montant de 300 millions par an pour les années 2020 à 2022 cette ponction ne saurait se poursuivre au-delà sans remettre en cause la structure même de cet organe du paritarisme à la française et dont les interventions en faveur du logement des salariés de la rénovation urbaine de coeurs de ville où les effets générateur pour nos territoires et nos communes ne sont plus à prouver, sachant qu'il restera 350 millions d'euros au 31 décembre en réserve au FNAP dont 200 millions sont fléchés et 150 à disposition pour justement accompagner encore le FNAP pour ces raisons, et donc en supprimant le grand 3 de l'article 16 je vous propose de mobiliser directement le reliquat des réserves du FNAP à hauteur de 150 millions d'euros qui viendront ainsi compenser partiellement la perte de recettes de 300 millions en complément, les partenaires sociaux pourront par voie conventionnelle et ils le feront, si c'est le cas venir compléter ce montant par un montant exceptionnel au Fnac en 2023 à hauteur de 150 millions d'euros dans le cadre des négociations en cours avec messieurs les Ministres, Béchu et un sur la convention quinquennale 2023 2027, par la voix de la convention et du partenariat aujourd'hui l'argent de la d'Action Logement n'est pas encore l'argent de l'État, même si on le sait, Monsieur le Ministre, c'est quand même une intention qu'au travers de ce qui se passe avec l'Insee, et effectivement de l'emploi hé bien malheureusement, à force de demander Action logement de se substituer à l'État, on prend le risque de retirer l'argent du paritarisme. C'est un repli du premier monsieur le Président, effectivement, c'est l'idée de ne remplacer les 300 millions par 150 millions sachant comme je l'ai rappelé : il reste 150 millions 31 décembre 2022 non affectées en réserve au FNAP qui pourraient compléter ces 300 millions. Merci madame la présidente, monsieur le rapporteur. la problématique qu'a rappelé la présidente les tard je rendrai un avis de sagesse sur l'amendement 1637 et je demande le retrait sur le 1636. Merci monsieur le président, oui, dans le cadre du projet de loi de finances 2023, le gouvernement a décidé de reconduire, je dis bien reconduire une contribution d'Action Logement au profit du FNAP à hauteur de 300 millions d'euros. Moi, je le dis, c'est ce qui va permettre la production de nouveaux logements, la rénovation de logements aussi, je veux dire que cette contribution d'Action Logement service au FNAP est parfaitement soutenable, du point de vue de leur trésorerie, ils ont une trésorerie importante qui leur permettra de faire face à ses engagements, je veux rappeler par ailleurs que Action Logement dispose du flux annuel de à la participation des employeurs à l'effort de construction qui est assis sur la masse salariale qui augmente nettement qui va continuer à augmenter dans les années qui viennent, donc c'est un milliard 7 en 2021, ça continue à augmenter, puisque le chômage baisse, la masse salariale augmente qui disposent des retours des prêts financés avec ce cette participation pour un milliard 300 millions d'euros additionnel et je veux dire que si ça n'est pas Action Logement qui contribue, ça devrait être la contribution des bailleurs. ça devrait être la contribution des bailleurs à la CGLLS, les bailleurs, on leur demande beaucoup, ils ont les prix de l'énergie qui augmente. Ils doivent construire, ils doivent rénover les logements aussi,

Donc voilà, par la reconduction de cette contribution d'Action Logement au Fonds national d'aide à la Pierre et justifiée sur le fond, soutenable en termes financiers, du point de vue de leur trésorerie et de leur recettes qui vont continuer à augmenter dans les années à venir, parce qu'elles sont assises sur la masse salariale qui augmentent et donc dans ces conditions, avis défavorable sur l'ensemble des amendements. Bien Madame Estrosi Sassone. à l'article 16 qui effectivement contraint Action Logement à verser 300 millions d'euros au FNAP la suppression de l'article 16 ferais porter le poids financier sur l'intégralité pour les bailleurs sociaux, l'article 40 nous empêche malheureusement de faire en sorte que la charge aillent à l'État, Monsieur le Ministre, ce qui serait parfaitement légitime parce que le FNAP il peut être abondé par les bailleurs sociaux par l'État et par Action logement mais pour autant dans les amendements que propose la présidente Létard avec la réduction de la contribution d'Action Logement, cela réduirait de fait les moyens du FNAP et empêcherait surtout de mobiliser et l'année prochaine les reliquats existants pour la rénovation des logements sociaux ou encore pour l'augmentation de l'aide unitaire au logement dans un contexte de hausse des coûts pour autant je rejoins complètement Valérie Létard sur les dangers qui pèsent sur Action Logement, et plus particulièrement sur le financement d'Action Logement Action Logement, service qui est une filiale d'Action Logement qui collecte et qui distribue l'APEC pour être classé demain effectivement en organismes divers d'administration centrale cela menacerait sa capacité à financer tous les programmes de renouvellement urbain, les actions, coeur de ville à financer également la garantie Visale ou même le FNAP mais cela conduirait surtout à une scission du groupe paritaire l'état de fait, contrôlant étroitement la collecte et l'emploi de l'APEC, ce que nous pouvons accepter, du tout que non, du tout de soi qu'un organisme paritaire collectant une contribution pour partie volontaire des entreprises soit classé comme Hodac, j'ajoute que le secteur du logement dans la situation dans laquelle il se trouve Monsieur le Ministre, comme les collectivités territoriales ont un intérêt stratégique à ce que Action logement reste un acteur et un financeur autonome donc no danger le danger est là, mais pour autant dans la loi de finances, nous ne pouvons pas nous nous sommes démunis parlementaire et nous ne pouvons pas enlever cette ponction qui est faite sur Action Logement, parce que cela rejaillit et sur les bailleurs sociaux, maintenance, Monsieur le Ministre, il faut que vous nous donniez de véritables garanties sur l'avenir d'Action Logement. Merci madame Jasmin. Oui merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, les bailleurs sans grande difficulté aussi parce qu'il y a un trou d'un pays est très important, il faut le savoir, les conséquences de toutes les crises sanitaires, sociales que nous connaissons, hé bien, et d'ailleurs ont de gros soucis, d'autre part, la participation des entreprises à l'effort de construction, ce n'est pas pour rien, donc vous allez des tricoté quelque chose qui fonctionne, les entreprises collectent des fonds et le BTP va mal aujourd'hui, nous avons un parc immobilier vieillissant en très mauvais état et nous sommes unanimes à reconnaître qu'il y a beaucoup de travaux à réaliser, donc le BTP ne va pas bien, les carnets de commande sont vides et vous vous voulez-vous ponctionner là où on peut encore faire des choses pour réparer le pire parce que quand un immeuble s'effondre et qu'il y a des morts qu'est-ce que vous en pensez donc je crois qu'il faut mettre la raison 150 millions pour à aborder et pas 300 millions merci.

Si évidemment avec Dominique Estrosi nous partageons avec victoire mais avec beaucoup de gens ici la même volonté et la même nécessité qu'il y a à financer effectivement accélérer l'effort de production de logements sociaux, la réponse de monsieur le ministre, elle est vraiment pas satisfaisantes parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit si Action logement ne paie pas, on fera pas mais c'est pas possible. Hou hou et l'État, dont l'ambition d'avoir une solution pour chaque Français, que ce soit dans la rénovation ou la construction de logements on occulte l'État combien d'argent, mais l'État dans la rue 15 millions cette année, sur combien un milliard de a été demandée, Action logement pour venir abonder ANRU 500 millions de leur rue allant rue supplémentaire d'Action Logement Action Logement accompagne coeur de ville accompagne Visale mais à chaque fois qu'Action Logement est sollicité pour financer les politiques publiques de l'État à la place de l'État, c'est à chaque Europe donner un euros en moins pour le logement, puisque ce devrait être additionnel l'argent d'Action logement pour le logement des salariés, on veut des infirmières dans les hôpitaux à Paris comme en fait si on n'est plus capable de les loger, hé bien c'est ça le sujet aujourd'hui, ce sont des euros pour le logement en moins, alors il faut effectivement et Action logement est toujours été solidaire des politiques publiques de l'État, mais Monsieur le Ministre, vous le savez bien, l'État peut prendre toute sa place aujourd'hui dans l'amendement qui vous est proposé, on met pas en difficulté la situation 200 millions des réserves sont affectés à la rénovation thermique des logements de l'USH, il reste 150 millions disponibles, on peut mettre 150 millions dans le cadre de la convention quinquennale, sur le modèle du partenariat et de la négociation et non pris par l'État sans discussion c'est c'est un changement de paradigme de la de ces financements et si ce n'est pas suffisant, il y aura des pays allaient faire l'année prochaine et peut-être que l'État pourrait utilement apporter sa contribution à l'effort du logement en France, mais là on est en train de changer de paradigme mais on tu veux vraiment Action logement et on conforte le fait que l'argent d'Action Logement devient l'argent de l'État, c'est l'argent des salariés.

mais ce ministre ou décréter unilatéralement que les opérateurs du logement ont les moyens de supporter cette mesure soutenable, dites-vous, mais quand même, les opérateurs du logement, ces dernières années ont pris quelques mauvais coups, je pense aux bailleurs, je rappellerai la réforme des APL, par exemple, qui a réduit qui a contribué à réduire leur capacité financière de manière importante, je m'étale pas sur les besoins en logements dans ce pays qui sont toujours pas réglés les besoins en terme de rénovation de par rapport à la crise climatique, le coût des matériaux qui flambent le coût du foncier, voilà autant de raisons qui font qu'il faut maintenir effectivement les moyens consacrés au logement Merci Monsieur Savary. et notamment quand il y a des gestions paritaires et et qui implique les partenaires sociaux et on voit bien que quand il s'occupe justement d'organismes hé ben c'est c'est mieux géré que quand c'est l'État qui s'en occupe donc il faudrait peut-être cesser ces pratiques, hier soir, vous nous avions une discussion où vous disiez que compte tenu de l'absence de majorité, cela avait changé, vous étiez dans un travail co-constructif, donc il est important justement de de tenir compte de ce que disent notamment les sénateurs dans ce domaine-là, que ce soit la ponction dans les chambres d'agriculture dans les chambres des métiers d'art, Action logement et caetera et, plus largement, et c'est là où je voulais en venir, on donne pas à travers ses actions de garantie de confiance aux partenaires sociaux, monsieur le Ministre je vous alerte, vous allez perdre la conférence des partenaires sociaux, on l'a vu à travers le PLFSS Monsieur le Ministre, en ne retenant pas dans à travers le quart entre trois le deuxième 49 3 la suppression de la de la comment on appelle du recouvrement des cotisations sociales par l'argile Arco qui devrait être confiée à l'Urssaf, là aussi, c'était le moyen de donner aux partenaires sociaux un gage de confiance donc attention parce que derrière cela, vous serez bloqués dans les réformes et ça ne ça n'incite pas à gérer correctement quand vous savez derrière que les gains que vous allez créer vont être ponctionnés merci.

et je crois que pour les stats, ceux qui ont pris la parole, on ne avait pas trop bavarder par rapport aux ce problème-là, c'est vrai que on est devant un réel dilemme Monsieur le Ministre, l'État ponctionne et nous les parlementaires si on voulait agir. Notre honorable président de la commission des finances. Nous soulèverait le fameux article 40. Donc que faire. Vous décidez et nous on subit. Mais j'allais dire, on est un moment important, je rejoindrai ma ma collègue Dominique Estrosi. Faisons attention quand même. En prenant des décisions, a pas pénaliser le logement social, je crois que surtout nos ben, quelles que soient nos territoires, moi j'entends notamment certains et je fais partie de ceux des des élus qui sont favorables aux logements sociaux, mais donnant une image aussi positive à nos mères qui puisse se produire du logement social n'ayant des bailleurs, dynamique et qui des finances alors faisons attention à travers cet amendement de ne pas arrêter la production de logements sociaux dans notre pays. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à mon tour, et sans en rajouter, vu leur particulièrement avancé, je voudrais dire que cette ponction de 300 millions d'euros, est proprement insupportable pour les raisons indiquées tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur, sur tout ce qui a été dit, il est clair que dans un contexte d'effondrement de la construction neuve des Français qui qui qui peinent à se loger au plus près de leur lieu de travail sont dans l'attente, naturellement, de, de, d'une solution à leurs difficultés, moi très franchement, monsieur le ministre, si on peut comprendre que les 300 millions pose problème : il y a un amendement de repli tout à l'heure à à 150 millions je, je militerai vivement pour que cet amendement de repli puissent avoir une écoute favorable de votre part, j'ai compris que le président le rapporteur, pardon, donner un avis de sagesse, moi je fais cet appel également, pourquoi ne pas aller vers cet amendement de repli qui a au moins cet Avantage c'est d'ouvrir des perspectives effectivement et de respecter un petit peu ce que font les partenaires sociaux, Je serai bref notre groupe partage à 100 % ce qu'a dit la présidente, l'État n'ai rien à ajouter ponctionner dans les caisses des autres, une nouvelle fois et mettre à mal le logement alors que tant de personnes, tant de familles sont en souffrance, c'est juste inacceptable.

Non, simplement pour dire que j'espère très sincèrement que celles et ceux qui. On parlait d'absence de l'État devant ses responsabilités de désengagement de l'État, d'un État pas au rendez-vous de ses responsabilités seront présents dans ce même hémicycle dans la partie de de ce budget qu'on sera discuter l'abondement d'un milliard 200 millions d'euros que nous avons décidé, pour financer le bouclier énergétique pour les logements sociaux, la facture d'électricité, de gaz, l'augmentation, c'est l'État qui va la payer. vous ne pouvez pas dire qu'un état qui fut sa responsabilité qui n'est pas au rendez-vous quand nous relevons le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie à hauteur d'un milliard 200 millions d'euros pour accompagner les bailleurs sociaux pour les aider à payer leurs factures et pour prendre en charge et c'est l'État qui la prendra la facture d'électricité pour dire que ça n'a rien à voir, c'est en fait, on est dans un moment difficile où l'État est amené à mettre en place un bouclier tarifaire, de près de 50 milliards d'euros pour protéger les Français, ça impose de faire des choix qui sont toujours des choix difficiles, ça ne donne pas les marges à l'État pour faire tout ce que nous voudrions faire et cela implique qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui prennent leur part et qu'il soient mis à contribution, oui je l'assume et je le dis, moi, je le redis, on est dans une situation financière qui est contrainte, on a fait ce choix de reconduction de 300 millions d'euros si les amendements sont adoptés, qu'il n'y a pas de changement dans la navette, ce qui n'est pas mis par Action logement sera mis par les bailleurs sociaux, je le dis, je le dis et Madame Estrosi Sassone a dit et donc ce seront non mais je je je je je suis franc avec vous et sincère, je ne le ferais pas le gage sur ces amendements et donc s'ils sont adoptés, s'il n'y a pas de changement dans la navette parlementaire, les 150 ou 300 millions d'euros, dont on parle, ce seront les bailleurs sociaux qui les payeront et ce seront eux qui seront mis à contribution, je le dis, je pense que c'est important d'être non c'est de la transparence, c'est la transparence, donc avis défavorable.

vous ne répondez absolument pas à la question, la question de du du bouclier tarifaire sur sur l'énergie, pourquoi on est obligé de le mettre en place, c'est justement parce que on prend un retard considérable sur la rénovation thermique, donc je pense qu'il ne faut pas tout confondre et sur les objectifs de production de logements sociaux, je rappelle que Madame wagon avait fixé en 2021 à 250000 sur 2 ans, soit 125000 logements, on est à peine à 80000 livraisons, donc on voit bien qu'on a besoin de boosté considérablement et que si on n'avance pas dessus, on voit bien qu'on est en train de constituer les éléments d'une crise du logement et donc vous en serez clairement responsable. Bien, nous allons passer, nous allons passer au vote sur ces deux amendements donc le premier le 16 36 avec un double avis défavorable,

Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté

Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Je mets aux voix, l'article 17. Qui est pour l'article 17.

Merci monsieur le président, dans notre vie parlementaire il y a les grandes phrases les grands discours et il y a le budget alors l'audiovisuel public, que tout le monde loue et notamment le gouvernement, qui ne cesse de dire que c'est absolument nécessaire dans le climat actuel de fake News de de plateformes géantes sur le plan mondial, qui contrôle l'information hé bien lui, depuis 5 ans n'a cessé de baisser ce budget, ce que pour Radio France, qui a fait des performances que tout le monde loue aussi il y a eu 340 emplois en moins et 60 millions d'euros en moins au budget sur la période 2018, 2022, et pour ce qui est le de France Télévisions ces 454 millions en moins et 847 emplois au moins, budget 2017, budget 2022, aujourd'hui on nous dit : mais ça y est, et le gouvernement fait un effort, alors comme je pose tout le temps, un amendement puisqu'il n'en fait pas, je me suis dit ben peut-être cette année, je vais pas en déposer puisque il fait un effort, hé bien non, il augmente, mais 2 fois moins que l'inflation, donc la baisse continue mais il va continuer à claironner qu'il a augmenté le budget de l'audiovisuel public et je le dis, monsieur le Ministre, vraiment, si on ne comprend pas, aujourd'hui, que c'est un enjeu pour notre société, cette question de l'information de la création culturelle, de l'audiovisuel, à un moment donné où on est inondé d'images qui viennent de n'importe tout n'importe où mais aussi de plateforme américaines ou étrangères ou chinoises qui formate l'opinion qui formatent les modèles culturels, alors on n'a pas compris comment préserver notre société y compris quand il y a de tels défis économiques et sociaux, un tel KO à la montée des extrêmes dans le monde.

Bien, je ne vais pas chercher à argumenter plus parce que ni le rapporteur d'ailleurs et encore moins le ministre non la décence de dire pourquoi ils sont défavorables. et je pense pas qu'on aille inondé le débat de cet enjeu de l'information sur des heures et des journées de débats sur le budget, mais je le répète si ici on considère et si, au gouvernement, on considère que là il y a un vrai enjeu de société, on se permet d'en dire un peu plus que défavorable je, je, je ne vais pas argumenter plus je sais que le gouvernement veut dire on continue comme avant, mais je le dis, quand on arrivera à ces grands états généraux de l'information que Emmanuel Macron a annoncé qu'on Vienne pas me dire que le gouvernement a pris la mesure de la chose parce que c'est dans les Budgets qu'on prend la mesure de la chose. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, monsieur Assouline le le compte de concours financiers pour l'audiovisuel public en 2023 le montant par des plans d'affaires des sociétés d'audiovisuel public il y a eu un travail extrêmement enfin qui a été fait avec les sociétés d'audiovisuel public pour qualifier les besoins, notamment en terme d'inflation, l'inflation ne s'applique pas de manière forfaitaire sur l'intégralité du budget de l'audiovisuel public sur certains postes l'énergie bien sur l'informatique sur quelques sur sur sur des postes identifiez vous avez une inflation qui s'applique, on a fait ce travail avec les sociétés d'audiovisuel public, poste de dépense par poste de dépenses pour qualifier celles qui sont en hein impacté par l'inflation et on en a tenu compte dans la dotation. Budgétaire qui est prévu, on n'a pas uniquement tenu compte de l'inflation, puisque votre amendement ne porte que sur l'inflation, mais on a aussi tenu compte du glissement de la masse salariale, on a tenu compte des dépenses engagées de la compensation des effets fiscaux induit par la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, parce que vous savez, vous êtes un spécialiste du sujet, qu'y compris en matière de taxe sur les salaires, il y avait des impacts tout ça, on en a tenu compte, ce qui fait que vous avez une dotation à l'audiovisuel public qui augmente de 114 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2022 donc votre volonté est satisfaite puisqu'on a tenu compte, via les plans d'affaires des entreprises de l'impact de l'inflation sur leurs dépenses. Bien, nous allons passer, nous allons passer au vote sur cet amendement. Avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous passons au vote sur l'article 18 qui est pour.

Donc, après l'article dix-huit l'amendement 1000 vingt-six monsieur Assouline. Oui, puisque le ministre m'a répondu : après ma réponse, je vais quand même lui dire que non, le budget de l'audiovisuel, cette année, j'ai remarqué qu'il avait augmenté, mais de un peu plus de 100 millions mais il a baissé de 462 565 millions pour Radio France et France Télévisions dans les 4 dernières années, et c'est pas dû cumuler puisque chaque année, ça veut dire que par rapport à 2018 il y a au moins, c'est 500 millions donc on ne retrouve pas rien, c'est pas seulement l'inflation, c'est mon amendement qui était modéré pour au moins dire que cette année ça doit rattraper l'inflation tous les responsables de l'audiovisuel public, c'est que, avec ce qu'ils ont aujourd'hui peut le faire que le minimum et le minimum, c'est laisser encore des parts de marché et être attaqué par les grandes plateformes je vous donne un exemple France Télévisions ne peut plus résister aux offres d'Amazon sur Roland Garros, donc même Roland-Garros ne sera plus sur le service public, à terme, parce que tous les droits augmentent et que les autres sont prédateurs en la matière, donc, pour faire le minimum, essayer de résister, peut-être, mais pour faire face aux impératifs tels que, aujourd'hui, ils sont devant nous, quand on voit la guerre en Ukraine qu'est-ce que ça signifie qu'moyen Poursuivre les choses vraiment et pour informer le monde et pour informer les citoyens face à la propagande de Poutine, donc je finis en vous disant que dans cet amendement, on va à la structure des choses vous avez supprimé le mode de financement pérenne. De l'audiovisuel, avec la redevance qui certes socialement été injuste et donc l'amendement que je propose là avec mon groupe, c'est un mode de financement pérenne par une redevance évolutive selon les les les moyens des ménages qui permet à 85 % des foyers de payer nettement moins que ce qu'on paye, avant de conclure, mais de garantir l'indépendance du financement que vous avez supprimé et en 2025, comme ce sera plus la TVA, il n'y a plus de financement prévu, on en reparlera. Merci je complète les propos de mon collègue David Assouline depuis la suppression de la contribution à l'audiovisuel public décidée au coeur de l'été, quelques semaines seulement après les élections présidentielles plusieurs propositions parlementaires ont émergé pour la remplacer, héritière de la taxe sur les postes de radio de 19133 l'existence d'une contribution affectée, a permis de développer par exemple les médias francophones, dont l'audience des bornes de nos frontières, c'est ce qu'a souligné le rapporteur Jean-Raymond Hugonet, qui souligne l'importance du rôle indispensable de France Médias Monde dans un monde troublé, nous avons proposé lors de la première loi de finances rectificatif 2 amendements, le 1er travailler avec l'économiste Julia KG qui rejoint celui de monsieur Assouline qui offre une solution à long terme, il prévoit de renforcer la progressivité du système qui était la principale limite de la C. P. en cria 4 taux correspondant à 4 tranches de revenus je compète sur la défense de leur l'amendement suivant l'autre amendement répond à l'urgence et souligne l'absence d'indexation de la fraction de TVA affectée à l'audiovisuel public défaut également relayé par notre rapporteur en commission culture, telle est l'esprit de ces deux amendements. Bien, merci, donc avis du rapporteur peut être sur les trois amendements, du coup, les 2 plus le suivant puisque Madame Marco la présenté en même temps. Ce sera 3 avis défavorable en tous les cas je je conclus par ces amendements qui a vraiment nécessité de se mettre au travail, on l'a dit, dans la foulée de la suppression de la redevance audiovisuelle, je crois qu'il y a pas de temps à perdre sinon je sens que les débats risquerait de se tendre il y a rien de tel que de vouloir amener une solution à la disparition de ressources hier pour financer le l'audiovisuel public, il y a 3 motifs hein je d'abord je suis. Pas spécialement favorable à la création de taxes notamment et je leur ai dit dans un contexte de forte inflation et de d'attention particulière portée au pouvoir d'achat des Français, pas, on n'achèterait pas pardon, avec l'adoption de cette taxe a des effets de seuil, voire à des injustices, je veux dire par là, pour les ménages dit dans les classes moyennes ça entraînerait des augmentations pour ces ménages et puis troisièmement, les effets de transfert, c'est le fait parfois d'avoir des cohabitations dans un même foyer, hé bien, dans ce cas-là, vous avez plusieurs personnes qui se trouvent pour un même service taxer ce qui ne me paraît pas non plus source de parfaite équité. Monsieur le ministre. Non, je veux dire à monsieur Assouline que les obligations d'investissement de France Télévisions dans les programmes dans leur contrat d'objectifs et de moyens, ces 420 millions d'euros la dotation qu'on leur verse pour leur permettre d'investir dans les programmes, c'est 440 millions d'euros, donc on leur verse plus que les obligations qu'ils ont dans leur programme d'objectifs et de moyens pour investir dans les programmes généreux avec les obligations d'investissement de France Télévisions pour le restant dans les programmes et il y a pas la disparition de plus belle la vie n'a pas entraîné de compensation pour pour autant je suis défavorable aux amendements, d'abord parce que je suis défavorable aux augmentations d'impôts et qu'en ce moment même 23 millions de Français devraient recevoir un avis de taxe de 138 euros et ils ne reçoivent, ils ne le reçoivent pas parce qu'on a supprimé la redevance et d'ailleurs la nouvelle redevance que vous proposez ne rapporterait même pas ce que rapportait l'ancienne contribution à l'audiovisuel public, ça sera donc une baisse massive du budget de l'audiovisuel public qu'on ne souhaite pas évidemment puisque ces 2 milliards de avec ces 2 milliards de avec

quand on déposera ce projet de loi alternative à votre mode de financement, mais il ne faut pas mentir, vous avez déjà menti sur d'autres sujets, et d'ailleurs on en reparlera peut-être pas seulement dans cette enceinte, mais il ne faut pas dire que les Français ne payent pas ce que vous avez proposé comme mode de financement, au contraire, c'est beaucoup plus injuste puisque c'est par la TVA, que tous les Français payent hors la loi que nous proposons alternative qui rejoint les différents scénarii qui ont été proposées à gauche est une loi qui permet que selon ses moyens on paye cette redevance et que 85 % des Français ne payer moins dans notre proposition, que ce qu'ils pouvaient payer avant et donc quelque chose de juste socialement et 2 progressif et la TVA, c'est l'inverse de l'impôt juste et progressif, donc arrêtez de dire ça, vous avez privé le budget de l'état d'une somme assez grande et vous arrêtez pas de nous dire qu'il y a pas d'argent pour ci, pour ça, pour le logement la la transition énergétique pour les transports avec ça, il y a pas d'argent, sauf que vous avez décidé de vous priver de cet argent, il y avait aucune manifestation dans le pays pour vous demander la suppression de la redevance, je ne crois pas, hein, par contre, ils vous demandent l'augmentation des salaires.

celle du savoir partager de l'information et de l'Intelligence ne se construira pas en livrant nos écrans à l'appétit dévorant des Gafam et des géants du numérique dont on connaît d'ailleurs les stratégies fiscales douteuses et ce qui permettrait de retrouver quelques sous pour financer notre système audiovisuel ça dépendra aussi de notre capacité de donner les moyens de répondre à la promesse de notre service public de l'audiovisuel Informer cultiver divertir. Ensuite, monsieur dessus. Oui, c'est un amendement qui propose de diversifier les sources de revenus pour l'audiovisuel public pour ne pas mettre tous les oeufs le le visuel dans le même panier de la ménagère ne pas ne pas dépendre que du bon vouloir de l'État, donc nous souhaitons faire contribuer, ça a été dit, les plateformes de contenus vidéo à la demande, mais plutôt que de mettre en place une nouvelle usine à gaz, nous proposons un dispositif assez simple puisqu'il s'appuie sur la taxe existante soit diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels sans créer de nouveaux prélèvements, nous proposons de renforcer le produit de cette taxe, en faisant passer le taux de 5 et demi à 10 % pour le contenu des plateformes en ligne, nous souhaitons en exclure les loueurs de films évidemment puisque la leur activité est loin d'être florissantes ne voulait pas pénaliser les restants la moitié du rendement de cette taxe serait affectée à l'audiovisuel public à côté et à côté du Centre national du cinéma et de l'image animée sont bénéficiaires actuels, c'est pas plateformes numériques agissent dans le domaine de l'audiovisuel en diffusant du contenu, elles doivent donc contribuer à l'écosystème qui les fait vivre. Monsieur le rapporteur. C'est marrant. Retrait pour le 824 2 éléments d'appréciation en doublant le taux pour en orienter la moitié du produit vers l'audiovisuel public, finalement ça reviendrait à dénaturer l'intention initiale du législateur et puis, il y aurait comme un paradoxe à faire participer des plateformes au financement de viser le public et donc des plateformes que le secteur public possède ou auxquels il participe et nous en avons quelques-unes en France sur le 903 jeux préciser que la taxe ne vise pas uniquement YouTube n'explique s'mais qui a également des plateformes françaises et, deuxièmement, une question de un problème de rendement puisque, avec un taux majoré de 10 % ça fait une recette de l'ordre de 90 millions d'euros, c'est une somme inférieure aux besoins de financement de l'INA je redis à nouveau, j'appelle le gouvernement à engager la réforme du financement du de l'audiovisuel public. Monsieur le Ministre défavorable, donc je soumets les amendements au voit avec un double avis défavorable, 800 vingt-quatre Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté le 903 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté ensuite l'amendement 58 madame Darcos. Merci monsieur le président, la loi de finances 2 pour 2020 harmoniser le taux des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée, en créant un taux unique de 5 15 en lieu et place du taux de 5,65 % pour la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs et du taux de 2 % pour la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels le présent amendement vise à prévoir un seuil de déclenchement de la taxe pour les éditeurs de services de vidéo à la demande, réalisant plus d'un 1000000 d'euros de chiffre d'affaires, à l'instar de celui qui existe pour la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs 10 millions d'euros cet abattement permettra d'atténuer l'impact considérable de l'augmentation du taux de la taxe 160 157 5 % % en intervenu en 2020 sur les acteurs du marché de la vidéo à la demande en s'inspirant du seuil retenu pour le conventionnement d'un service avec la comme il s'agit ainsi d'appliquer une forme d'abattement qui existent pour les chaînes linéaires à l'heure où la consommation se répartit entre ces 2 modes de visionnage une pluralité d'offres est indispensable au consommateur dans un paysage déjà largement concentré entre les mains de plateforme internationale. Demande de retrait Monsieur le Ministre, même avis vous le maintenez Madame Darcos oui, donc je le soumets aux voix qui est favorable à cet amendement.

Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté,

à hauteur de 26 millions et une contribution des organismes de gestion collective des droits qui fait qui font 1 virgule 5 millions d'euros, c'est trop peu, alors bien sûr, l'État a contribué à hauteur de 200 millions d'euros durant les 2 années de la crise Covid mais ce soutien a été ponctuel et n'a pas vocation à se poursuivent donc, nous posons la question de la contribution des nouveaux acteurs de la filière musicale numérique les plateformes comme Spotify ou 10 heures qui propose la diffusion de contenu musical dématérialisé, nous proposons de faire payer une taxe à hauteur de 1 virgule 5 pour alors à ceux qui s'inquiéteraient que cet amendement marche sur les plates-bandes de la mission de notre collègue, bargeton, qui a une mission pour le financement de la musique nous considérons au contraire que si nous assisterons cette taxe dès maintenant la mission pourra justement en dresser une première évaluation et des le législateur a corrigé le Tir pour l'année prochaine.

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté ensuite l'amendement 676 qu'présente. Madame Gosselin.

Il a retiré, donc je vais mettre aux voix l'article 19 qui est pour l'article 19. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté l'article auvent même vote. Le vote, l'article 21 même vote. Même votre l'article 22 même vote. Et la. Sur l'article 23, un amendement du gouvernement.

Oui merci monsieur le président Monsieur ne sera pas trop cher, cher collègue, cet amendement revient sur la décision de supprimer au bénéfice des communes de la part communale et de la part départementale concernant la redevance sur les concessions hydroélectriques puisque cette redevance et les calculé sur une parité entre 50 % pour l'État 50 % pour les territoires répartis entre départements et régions, et effectivement c'est notamment de mort redonne la possibilité, comme c'est fait partie des règles je dirais de cette répartition puisque ça concerne correspond quand même, soit 100 millions donc 66 millions pour la part départementale et 33 millions pour la part communale. Avis du rapporteur. j'ai eu l'occasion de le dire, j'y suis athée assez attachés au maintien de recettes des collectivités territoriales mais je juste dans le même temps, donner les de manière à ce qu'on puisse se prononcer de manière la plus objective possible la redevance qui est visée par l'article 24 bis concerne en fait 20 départements et un peu plus de 150 communes. Ce qui est proposé par un produit où on avait auparavant l'an passé 9 millions d'euros de recettes à partager aujourd'hui c'est plus de 200 millions 20 départements 150 communes, il est proposé, qui a un écrêtement sur cette somme, à part au-delà de 100 millions d'euros qui restent aux communes, le reste allant à l'État. Une proposition de sagesse. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, effectivement, vous avez un peu plus d'une centaine de collectivités qui ont des recettes spécifiques liées à des concessions hydroélectriques en 2022, le montant des deux. Ces recettes est passé de 10 millions d'euros à 80 millions d'euros fois et il devrait être de 200 millions d'euros l'an prochain, du fait de l'augmentation des prix de l'électricité sur le marché, il y a donc une forme d'effet d'aubaine, que ces recettes, d'ailleurs, d'abord il y a pas de perte de recettes, puisque les recettes continueront à dynamique pour les collectivités concernées on ne propose pas que les recettes supplémentaires à l'État, mais elles vont venir financer en partie et en petite partie puisqu'il coûte 50 milliards d'euros, le bouclier énergétique dont vont bénéficier tous les Français et toutes les collectivités avec le filet de sécurité ce que vous avez voté on laisse la recette continue à progresser et nettement aux collectivités locales concernées 130 collectivités locales concernées jusqu'à 100 millions d'euros, je rappelle que c'était 10 millions d'euros quand même avant l'effet d'aubaine que constitue la spéculation et le reste ira financer le filet de sécurité dont bénéficient toutes les collectivités locales qui n'ont pas la chance d'avoir une concession hydroélectrique qui leur permettent d'avoir cette entre guillemets, effet d'aubaine au moment de la crise énergétique, donc avis défavorable sur l'amendement. Donc un avis défavorable du gouvernement Monsieur Gremillet. Oui, monsieur le président moi je, je vais maintenir cet amendement pour une simple raison, c'est la réalité des territoires sur tel territoire il y a de l'hydro-sur telle autre territoire il y aura de l'éolien sur d'autres territoires, il y aura du photovoltaïque sur un autre territoire, c'est, c'est la réalité de de la France de de cette richesse, il y a eu des investissements sur l'hydroélectricité sur certains territoires, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, Monsieur le Ministre, il y a pas d'effet d'aubaine, c'est la réalité de ce qu'on est en train de vivre, c'est la même chose pour les autres énergies et aujourd'hui privées les communes de de cela a privé cela aussi au niveau des départements quand je vous entends ce renversement les phénomènes il est autant pour le l'État puisque vous allez grâce à la situation du marché avoir 100 millions de plus donc je ne vois pas au nom de quoi on priverait de cette situation de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui à la fois les départements et les régions, je maintiens ce cet amendement.

nous notre logique, c'est de dire on veut capter ce qui dépasse les coûts de production, une éventuelle augmentation des coûts de production et une marge raisonnable, ce qui est lié à la spéculation et à l'inflation des prix de l'électricité pour le coup, on le prend pour financer le bouclier de tous les Français est-ce que les 130 communes qui ont une concession hydroélectriques ont vu leurs charges liées à ces concessions hydroélectriques augmenter pour autant, il y a des recettes qui augmentent parce qu'il y a une spéculation et une inflation sur les prix de l'électricité, ce qu'on dit, c'est qu'une grande partie du fruit de cette inflation va continuer à aller à ces communes, c'est 130 communes concernées mais que le reste va aller au filet de sécurité, qui va financer toutes les collectivités, ça me semble être assez juste et assez justifiée sur le fond.

Bien, donc nous allons passer au vote sur cet amendement, qui est favorable à cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Maintenant, sur l'article 24 bis qui est, qui est pour l'article 24 bis.

qui nuisent et entrave l'attractivité des territoires ruraux, elle favorise largement le départ de nombreux professionnels de santé de zones rurales pour se rendent dans les ZFU ainsi concrètement le professionnel de soins, désireux de s'installer dans une zone sur-dotée ne pourra jamais bénéficié des avantages ZFU tandis que celui, désireux de s'installer dans une zone normale, voire sous-dotées sera éligible à l'aide. Merci, avis du rapporteur. qui lierait le fait qu'il y a de nombreux départs de professionnels de Santos, zones rurales pour se rendre dans les ZFU puisqu'en fait il y a qu'une centaine de ZFU qui concerne un 1000000 et demi d'habitants je suis également sceptique sur la portée de l'amendement, d'abord parce qu'il y a des conventions avec les professionnels, et vous allez avoir, on aura du mal à pourvoir, on aurait du mal à pouvoir couvrir l'ensemble des professionnels de santé sur le la question des des zones sous-dotées, enfin l'amendement soulève la question finalement de la pertinence du jaune, du zonage de l'efficacité des incitations fiscales et sociales et des éventuels effets pervers

Bien, cher collègue, la parole est à Rémi Féraud, pour une mise au point au sujet d'un vote. Merci monsieur le président je veux faire une rectification de vote au nom de notre collègue collègue Rachid Temal sur les scrutins publics 66 et 67 hier puisque ils souhaitaient voter contre sur ces 2 scrutins. Bien donné de votre mise au point, chers collègue elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés avant de suspendre la séance, je donne la parole au président rénale.

nous y sommes arrivés avec des les efforts, les efforts collectifs mais ce que je me suis permis d'encourager régulièrement, je voudrais dire simplement que le dernier amendement de monsieur sera évidemment vu tout à l'heure, puisque c'est un amendement sur l'article d'équilibre je voudrais dire aux membres de la commission des finances que nous nous retrouverons du coup à à quatorze heures trente non pas en séance mais en commission pour examiner cet article d'équilibre qui entre temps vous sera proposé par le gouvernement, et nous nous retrouverons, mais le président me le redire donc un quart d'heure plus tard en séance. Bien, merci, donc je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 14 heures 50 pour l'examen de l'article d'équilibre du projet de loi de finances pour 2023 suivie par les explications de vote et le scrutin de public ordinaire de droit sur la première partie, la séance est suspendue.